La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du mercredi 29 mai 2019 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé

Madame la présidente, supérieur, monsieur le rapporteur, messieurs les rapporteurs pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, c'est avec humilité, mais détermination, que j'aborde, cette semaine, l'examen du projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé. Je mesure pleinement les attentes dans vos territoires et l'exigence particulière, dans cet hémicycle, d'une réponse aux inquiétudes des citoyens et des élus. cette exigence, c'est d'abord et avant tout permettre à notre système de santé de tenir, demain, les promesses qu'il a toujours tenues. C'est l'enjeu de ce projet de loi et c'est ce que les Français demandent avec une insistance parfaitement justifiée.

Nous n'avons pas le choix, il faut répondre à l'urgence, dans des territoires qui se sentent abandonnés, et anticiper le déclin démographique. Les défis structurels auxquels nous sommes confrontés sont le résultat de plusieurs facteurs, et je sais que nous partageons les mêmes constats. Un exemple me semble bien illustrer cet échec collectif de 1991 à 2000, moins de 4 000 médecins ont été formés chaque année. Nous payons aujourd'hui au prix fort ce manque d'anticipation, à l'heure où le vieillissement de la population et l'augmentation du nombre de maladies chroniques deviennent des phénomènes de très grande envergure. Dans un contexte d'inégalités grandissantes dans l'accès aux soins et de mutations démographiques majeures, la transformation de notre système de santé n'était pas une option, c'était une nécessité absolue. Nous proposons donc un changement de paradigme, qui est aussi un changement de culture, en raisonnant désormais autour de deux axes le temps médical accessible ou disponible, qui consiste à permettre aux médecins de faire ce pour quoi ils sont les mieux qualifiés, et, d'autre part, le décloisonnement, pour que l'exercice isolé devienne l'exception et l'exercice coordonné la norme. Notre ambition- et je sais que nous la partageons tous -consiste à transformer notre système de santé dans son ensemble ; qu'il s'agisse des modes d'organisation, du financement, la formation ou des conditions d'exercice des professionnels, nous ne devons négliger aucun moyen pour garantir et améliorer l'accès à des soins de qualité pour tous, dans tous les territoires. C'est la vocation de ce projet de loi que d'être l'un des instruments de cette transformation globale. D'autres leviers- réglementaires, conventionnels, financiers, mais aussi d'animation territoriale et d'appui aux acteurs -viendront prolonger la loi. Je pense en particulier

En matière d'organisation, je pense au développement des communautés professionnelles territoriales de santé, qui conduiront à une meilleure coordination des professionnels de santé pour améliorer l'accès aux soins de la population dans les territoires. Je cherche à rassembler tous les acteurs autour de notre stratégie, et cette approche porte ses fruits puisque, hier, un premier syndicat de médecins généralistes a apporté son soutien à nos propositions, en annonçant qu'il signerait avec l'assurance maladie la convention sur les assistants médicaux et les communautés professionnelles territoriales de santé. C'est avec cet élan et cette adhésion que nous répondrons à la question de l'accès aux soins.

La Paces cédera la place à un système qui demeurera sélectif et exigeant, mais qui fera une meilleure place aux compétences, au projet professionnel et à la qualité de vie des étudiants. En développant les passerelles entrantes, la diversité des profils sera également privilégiée. Le deuxième cycle des études médicales sera rénové, avec la suppression des épreuves classantes nationales. Il s'agira de créer une procédure d'orientation qui prenne en compte les connaissances, mais aussi les compétences cliniques et relationnelles, et qui soit respectueuse des projets professionnels des futurs médecins. Frédérique Vidal, avec qui je porte les premiers articles de ce projet de loi, vous précisera les détails de ces deux mesures dans quelques instants. Le titre II s'attache à structurer des collectifs de soins de proximité dans les territoires. La création de projets territoriaux de santé doit aider à mettre en cohérence les initiatives de tous les acteurs des territoires, quel que soit leur statut- libéral, en exercice regroupé ou coordonné, hospitalier, du secteur social ou médico-social, public ou privé -, en associant évidemment les élus et les usagers. Ce sont ces projets territoriaux qui formalisent le décloisonnement, pierre angulaire du plan Ma santé 2022. Le statut des hôpitaux de proximité sera revu. Nous voulons que ces derniers soient mieux adaptés aux soins du quotidien et ouverts sur la ville et le médico-social. Les missions socles ont été inscrites dans la loi, tandis que les modalités de financement seront définies par les prochaines lois de financement de la sécurité sociale. Je profite d'être devant vous cet après-midi pour le rappeler : il n'y a pas de carte hospitalière cachée. Au contraire, les hôpitaux de proximité sont une chance pour les territoires, nous allons y investir des moyens financiers importants et, avec la gradation des soins et les consultations avancées, nous assurons à tous nos concitoyens des soins de qualité en proximité. Un chapitre du projet de loi est également consacré à l'acte II des groupements hospitaliers de territoire. Nous estimons que le projet médical doit désormais être le centre de gravité de ces groupements. La gestion des ressources humaines médicales sera mutualisée, et la gouvernance médicale sera adaptée et renforcée en conséquence dans les établissements de santé. Un nouvel article du projet de loi, introduit à l'Assemblée nationale, offre également la possibilité aux professionnels paramédicaux de la filière de rééducation de cumuler une activité libérale, en ville, avec une activité publique, à l'hôpital cette mesure devrait permettre de faciliter l'exercice des kinésithérapeutes et des orthophonistes dans les hôpitaux. Plus largement, l'examen à l'Assemblée nationale a conduit à modifier le périmètre de compétences de certaines professions de santé. Je pense en particulier à la délivrance, par les pharmaciens, de médicaments sous prescription médicale obligatoire, et à l'ouverture aux infirmiers de la possibilité d'adapter des prescriptions et de prescrire certains produits en vente libre. Derniers pivots du projet de loi, qui sont aussi des conditions de notre réussite collective : l'innovation et le numérique. Notre ambition est de redonner à la France les moyens d'être en pointe sur ces sujets. Nous inscrivons ainsi dans la loi le Health Data Hub, qui favorisera l'utilisation et l'exploitation des données de santé dans les domaines de la recherche, du pilotage du système de santé et de l'information des patients. Nous créons aussi l'espace numérique de santé, un compte personnel en ligne, qui permettra à chacun d'accéder au dossier médical partagé, à des applications sécurisées et à des informations de santé. La dématérialisation des pratiques passera aussi par le renforcement de la télésanté. La création du télésoin permettra à des paramédicaux et à des pharmaciens de réaliser certains actes à distance, et cela ouvrira de nouvelles opportunités sur les territoires, dans des filières sous-dotées comme en orthophonie. J'aimerais enfin partager avec vous une conviction : la politique que nous conduisons dans le champ de la santé ne peut se faire sans nouer une relation de confiance durable avec les élus. J'ai évoqué la nécessité du décloisonnement entre les professionnels de santé ; ce décloisonnement, il faut aussi le mettre en oeuvre entre l'État, ses services déconcentrés, les opérateurs et les collectivités territoriales. Pour construire le système de santé de demain, il ne faut pas de décision imposée d'en haut. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, messieurs les rapporteurs comme ministre, notre stratégie et ce projet de loi sont la meilleure réponse. Représentants des territoires et témoins privilégiés de la détresse de nos concitoyens,

Je le crois fondamentalement, un pays qui sait soigner est un pays qui peut guérir. La parole

les perspectives de long terme qui adapteront celui-ci aux évolutions épidémiologiques et préserveront notre modèle social. Cela nécessite que les professionnels de santé, dont les médecins, travaillent autrement. La coopération de différents professionnels, du patient et de l'entourage de celui-ci, au service du projet du patient, sera un élément déterminant de la qualité et de l'efficience du système de soins. L'évolution des connaissances et des techniques continuera de transformer profondément et rapidement les métiers des professionnels de santé. L'intelligence artificielle au service du diagnostic, la génomique au service de la personnalisation des traitements, la télémédecine pour mettre à disposition de tous nos concitoyens l'expertise la plus pointue : voilà trois exemples, issus de notre capacité de recherche et d'innovation, qui induiront des évolutions majeures des métiers de la santé. Dans tous les domaines d'activité, il faut, dès que l'on aperçoit l'horizon d'un changement majeur des compétences mobilisées, adapter sans délai le système de formation, premier facteur déterminant notre avenir, et donc notre première responsabilité vis-à-vis des générations futures. C'est pour ces raisons que les deux premiers articles de ce projet de loi vous proposent une transformation majeure des études de santé et, plus spécifiquement, des études de médecine.

Le premier article du texte supprime le et la Paces, que le Président de la République qualifiait, en septembre dernier, d'« acronyme funeste menant de bons lycéens à l'échec En quelques mots, il s'agit, avec ces deux dispositions, de faire vivre, dans la formation des médecins, tous les principes qui ont sous-tendu la loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation promouvoir la réussite des étudiants- tous les étudiants -, en diversifiant les profils des futurs médecins et en offrant une pluralité de voie d'accès aux filières de santé. Aujourd'hui, plus de 40 000 étudiants s'inscrivent chaque année en Paces ; ce sont de bons lycéens, mais plus d'un tiers d'entre eux reprennent à zéro, après deux années vécues comme deux échecs, un cursus, et quelques-uns, parmi les plus fragiles, en sont durablement brisés. D'autres, anticipant ce risque, et ne disposant pas du soutien familial et social pour le prendre, n'osent même pas formuler ce projet ; cette autocensure participe à la reproduction sociale qui caractérise ces études. Cette situation n'est pas compatible avec notre volonté que chaque jeune, d'où qu'il vienne, ait les mêmes chances de mettre ses talents au service de la société tout entière. Demain, un lycéen pourra commencer ses études supérieures dans une diversité de cursus. Dans ce cadre, il aura tous les atouts pour réussir et choisir, s'il le souhaite, de présenter sa candidature pour se lancer dans les études de santé. Celles-ci resteront évidemment sélectives ; l'excellence académique mais aussi d'autres compétences, utiles à ce métier, dans lequel la communication interpersonnelle tient tant de place, permettront aux candidats d'accéder aux filières de santé. Le travail réalisé par les parlementaires a permis d'affiner ce premier article, de préciser dans la loi les grands principes qui doivent organiser l'admission des étudiants, dont celui de la nécessaire diversité des voies d'accès, de définir les organisations qui devront être fixées par les textes réglementaires et de maintenir une marge importante d'autonomie des acteurs locaux. Les concertations que nous conduisons avec les acteurs sont extrêmement constructives. Nos universités ont préparé les parcours de licence permettant d'associer des contenus de santé à d'autres disciplines, et nous devons les aider à mettre ces évolutions en oeuvre dès 2020, pour faire cesser le gâchis de la Paces. Nos concitoyens nous l'ont répété avec force au cours des derniers mois leurs élus sont les premiers auxquels sont adressés leurs messages, leurs demandes, leurs colères et parfois leurs détresses. Agnès Buzyn et moi-même l'entendons sans cesse lors de nos déplacements.

Pour autant, nous devons aussi la vérité à nos concitoyens. Aucune mesure ne permettra d'augmenter dès demain le nombre de médecins formés, et l'accès aux soins doit être amélioré par d'autres moyens ; ceux-ci figurent dans ce projet de loi. dit, les études de médecine et, plus généralement, les études de tous les professionnels de santé doivent être repensées, avec pour souci constant de servir à terme les besoins de santé de la population et de former les professionnels dont nous avons besoin. Les parlementaires ont proposé plusieurs évolutions du texte en ce sens, et nous serons bien entendu heureuses d'émettre un avis favorable sur celles-ci. Oui, bien sûr, comme l'a proposé le sénateur Lafon, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, l'organisation des études de médecine doit favoriser une répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire, au regard des besoins de santé. Ce point est si important qu'il mérite de figurer dans le projet de loi, le concept de responsabilité sociale des facultés de santé. Le deuxième article exprime, plus tard dans les études médicales, notre ambition de concilier exigence, bienveillance et ouverture. Aujourd'hui, les études de médecine représentent un saut d'obstacles ne convenant qu'à un type d'intelligence. L'étudiant, sélectionné par des questionnaires à choix multiples en Paces, accède ensuite à telle ou telle spécialité en fonction de sa capacité à mémoriser une grande quantité d'informations et à cocher des cases. Les qualités de synthèse, de décision en situation d'incertitude ou, plus simplement, la capacité à conduire un entretien ou un examen clinique sont peu évaluées et, finalement, ne comptent pas dans l'orientation, pas plus que le fait de s'être impliqué dans un travail de recherche ou d'avoir une expérience internationale. Est-ce bien cela que nous voulons pour nos futurs médecins ? En tout cas, eux nous disent clairement le contraire ; ils ne veulent plus de ce modèle dans lequel le bachotage intensif leur fait perdre le sens même de ce qui les avait conduits à s'engager dans cette voie. Nous vous proposons donc de mettre fin à cette situation, de diversifier les critères d'évaluation des étudiants et de construire des parcours multiples, en perspective de l'internat du troisième cycle. Je suis convaincue que, ainsi mieux formés, ces étudiants nous soigneront mieux. L'organisation du deuxième cycle devra également tenir la promesse de former les professionnels dont les territoires ont besoin. résolument choisi de privilégier la découverte de tous les modes d'exercice, la diversité des terrains de stage et la qualité de l'encadrement pédagogique plutôt que les mesures coercitives. Envoyer un étudiant faire un stage à un endroit où il serait mal encadré n'est pas le meilleur moyen de susciter son intérêt pour l'exercice dans ce territoire. Gageons qu'il sera plus efficace de former à la maîtrise de stage des professionnels regroupés

Dans le même temps, l'organisation du deuxième cycle et les mesures d'accompagnement, par exemple de la mobilité, mises en place par l'État et par les collectivités locales, doivent favoriser des stages dans tous les territoires. C'est ensemble- État et collectivités, enseignants et étudiants -que nous relèverons ce défi. Voilà en quelques mots la vision du Gouvernement sur cet aspect spécifique du texte ; deux articles pour transformer les études de santé, deux articles dont les lignes de force sont la réussite et l'épanouissement des étudiants, la diversité des trajectoires et des talents, la garantie de la compétence des professionnels au service de tous les territoires. Je me tiens naturellement à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. La parole est à M.

Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, nous engageons l'examen d'un projet de loi dont l'intitulé est riche de promesses : il entend réformer l'organisation de notre système de santé, mais aussi le transformer. cette ambition, comme nous avons partagé le diagnostic posé à l'issue de la stratégie de transformation de notre système de santé, dont chacun a reconnu la justesse. Cette concertation a fait émerger une volonté commune des acteurs de refonder un modèle décrit, à juste titre, comme à bout de souffle. Le projet de loi qui nous est soumis présente des inflexions positives. La refonte attendue des études de santé permettra une sélection plus progressive des futurs professionnels médicaux et une diversification de leurs profils. Néanmoins,

Permettez-moi d'exprimer deux principaux regrets. Le premier tient au contenu même du projet de loi, qui s'apparente, à bien des égards, à un cadre général d'orientations. Le renvoi très large à des ordonnances ou décrets, sur le contenu desquels nous avons encore peu d'éclairages précis, laisse beaucoup d'interrogations en suspens. Nous comprenons la nécessité de poursuivre la concertation, mais le calendrier retenu pour l'examen de ce texte aboutit, nous le déplorons, à appauvrir le débat parlementaire. Sur des sujets majeurs pour les territoires, comme les hôpitaux de proximité ou les évolutions de la carte hospitalière, le débat aurait été plus serein s'il avait pu porter sur un modèle plus abouti. La commission n'a toutefois pas souhaité faire obstacle à l'avancée des réformes, mais elle attend que nos échanges permettent d'en affiner les contours. À côté de ce sentiment d'inachevé, mon second regret touche à ce que nous n'avons pas trouvé dans le texte. Ce projet de loi peut-il prétendre transformer notre système de santé sans évoquer ni sa gouvernance ni son financement ? Il me semble que nous ne pouvons plus ériger en priorité le décloisonnement des acteurs de santé sans revoir les contours d'un pilotage national qui contribue, en lui-même, à accentuer des logiques de silo. De même, nous voyons que toute tentative pour adapter les moyens d'action aux besoins des territoires se heurte à des limites dans une administration de la santé fortement centralisée. Je regrette que ce projet de loi ne pose pas les bases d'évolutions de fond sur ces sujets. J'aurais souhaité, mesdames les ministres, y retrouver le souffle des grandes réformes en santé, dans la lignée des ordonnances Debré ou même, à un degré moindre, de la loi HPST, qui avait rénové en profondeur la territorialisation des politiques de santé et la gouvernance hospitalière. L'ambition de ce texte réduit nos capacités d'initiative pour porter certains sujets. Je souhaite que nous poursuivions ensemble la réflexion, en particulier pour envisager, en matière de prise en charge des soins, le passage d'une architecture à double étage au principe d'un payeur unique. J'y vois un levier d'efficience, mais également un enjeu de lisibilité, et donc d'adhésion à notre modèle de sécurité sociale. Vous connaissez également, madame la ministre, mes réserves quant aux modes actuels de financement des investissements, notamment immobiliers, des établissements de santé je n'ai pu inscrire dans le projet de loi le principe d'une banque des investissements, mais je souhaiterais que votre ministère puisse approfondir la réflexion sur ce sujet crucial pour l'avenir des hôpitaux. en soit, la commission des affaires sociales a abordé l'examen du texte qui nous est présenté dans un esprit constructif. Ses apports ont été guidés par deux priorités : les territoires et l'ambition numérique. Sur le premier volet, nos concitoyens ont exprimé, lors du grand débat national, des attentes fortes à l'égard du système de santé. Le satisfecit sur la réforme des études de santé

et une sélection demeurera, selon des modalités certes nouvelles. Surtout, la réforme n'aura pas d'effet à court terme sur la démographie médicale, le n'ayant au demeurant pas de lien avec la répartition territoriale des praticiens. Sur le sujet sensible de la présence médicale dans nos territoires, nous savons qu'il n'existe pas de solution miracle. Je me réjouis que les échanges constructifs qui se sont poursuivis au sein de notre commission, associant différents groupes, puissent aboutir à proposer, au cours de nos débats, des évolutions utiles autant que pragmatiques. D'autres propositions adoptées par la commission visent à encourager les jeunes praticiens à un ancrage rapide au sein d'un territoire et auprès d'une patientèle : d'une part, une incitation fiscale forte à l'installation rapide au sortir des études, d'autre part, une limitation de l'exercice comme remplaçant. Une autre ligne directrice de nos travaux s'appuie sur la confiance dans les acteurs de terrain et dans les collectivités territoriales. Je reconnais que, en s'inscrivant dans la continuité de la loi Touraine, adoptée voilà juste trois ans, ce projet de loi, pour un pragmatisme bienvenu ; les acteurs commencent à peine, en effet, à se saisir des outils mis en place par cette loi, comme l'ont montré nos collègues Catherine Deroche, Véronique Guillotin et Yves Daudigny dans un premier bilan. Cela dit, si la commission a soutenu l'élaboration d'un projet territorial de santé comme levier du décloisonnement indispensable entre la ville, l'hôpital et le médico-social, je regrette que, une fois encore, on superpose et complexifie les outils. Veillons à ne pas décourager les porteurs de projets en gardant des dispositifs souples, sans céder à la tentation d'une hyperadministration de la santé. Suivant la même logique, la commission a privilégié les démarches de volontariat des établissements pour la poursuite de l'intégration au sein des groupements hospitaliers de territoire. Il me semble que l'hétérogénéité des situations actuelles ne doit pas conduire à imposer à tous un schéma homogène. Un autre axe d'évolution porte sur le lien entre l'État en région, à travers les agences régionales de santé, les ARS, et les élus du territoire. À mon sens, ce lien est aujourd'hui à repenser très largement. Et ce n'est pas en associant les parlementaires à des instances locales, en palliatif à la suppression du cumul des mandats, que nous y parviendrons. La commission a privilégié des mesures plus opérationnelles, avec un renforcement des prérogatives du conseil de surveillance des ARS et du poids des élus locaux en son sein. Elle a également consolidé, en adoptant des amendements du groupe socialiste, le rôle de pilotage stratégique des conseils de surveillance des hôpitaux. Sur la transformation numérique de notre système de santé, la commission a reconnu l'urgence d'agir en confirmant la mise en place d'une plateforme des données de santé et en rendant automatique l'ouverture d'un espace numérique de santé, levier de la coordination indispensable des parcours de soins. Parallèlement, elle a conforté les obligations en matière d'accessibilité pour nos concitoyens éloignés des usages numériques. pour ne pas prendre un retard qui serait ensuite impossible à rattraper, la commission a renforcé les exigences d'interopérabilité applicables au secteur en instituant un mécanisme de certification, accompagné d'instruments à visée incitative pour les éditeurs. Telles sont, madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, les orientations qui ont guidé notre commission des affaires sociales dans l'examen de ce projet de loi. Nous avons apporté des inflexions à un texte dont nous reconnaissons les apports tout en regrettant les limites. En définitive, ce sont les moyens accordés pour accompagner son déploiement qui signeront, ou non, la réussite de cette réforme, là où les précédentes lois ont échoué à répondre à l'urgence d'une refondation de notre système de santé. Nous y resterons évidemment attentifs. Je remercie nos collègues rapporteurs pour avis, Laurent Lafon et Jean-François Longeot, pour le travail qu'ils ont réalisé au sein de leurs commissions respectives et pour le regard complémentaire qu'ils ont porté sur ce texte, même si nous n'avons pas toujours été d'accord sur des sujets importants- et nous resterons en désaccord encore longtemps ... En conclusion, la commission des affaires sociales vous demandera d'adopter ce projet de loi, sous réserve des amendements qui contribueront encore à l'enrichir. La parole est à M.

Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, sur l'initiative de sa présidente, Mme Catherine Morin-Desailly, le bureau de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a décidé de rendre un avis sur ce texte, transmis au fond à la commission des affaires sociales, mais dont plusieurs dispositions intéressent la commission, et tout particulièrement les articles 1 à 2 qui traitent de la réforme des études de santé. Cette réforme, qui fait largement consensus, a recueilli l'aval de notre commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Nous avons notamment apprécié la méthode qui a prévalu et qui a permis de dégager un assez large consensus. Saluons ici la mission du professeur Jean-Paul Saint-André, les différentes expérimentations et concertations avec les professionnels de santé, la mise en place de véritables groupes de travail, les nombreuses contributions écrites et les auditions, organisées au Sénat, aux côtés des conférences des doyens de facultés de santé, de la conférence des présidents d'universités, ou encore des organisations représentatives des étudiants. Je tiens également à remercier M. le président et rapporteur, Alain Milon, mais aussi notre collègue Jean-François Longeot, rapporteur pour avis et, bien évidemment, Mme la présidente Catherine Morin-Desailly. Les inconvénients de la Paces à à l'entrée dans les études de santé et ceux des épreuves classantes nationales à l'entrée en troisième cycle des études de médecine ont été assez largement dénoncés. Avec un taux de réussite inférieur à 30 %, le système met en échec de très nombreux jeunes, pourtant excellents bacheliers. Le coût pour les familles, comme pour la Nation, est également lourd et excessif. La Paces est plus une année de sélection qu'une année de formation véritable. Les conditions d'études y sont peu satisfaisantes- amphithéâtres surchargés, quasi-absence de travaux dirigés ... Surtout, le recrutement se fait selon un profil type très stéréotypé, celui du bachelier scientifique, titulaire d'une mention très bien et issu des classes sociales les plus favorisées. Les expérimentations menées depuis 2013 et dont le nouveau dispositif s'inspire assez largement ont montré leur intérêt en termes de diversification des profils recrutés et d'instauration de parcours de réussite pour les étudiants. Notre commission s'est interrogée sur la précipitation avec laquelle la réforme de la Paces va être mise en oeuvre. Il nous semble peu réaliste de demander aux universités d'avoir élaboré toutes leurs nouvelles maquettes de formations dans moins de six mois. Si les universités se contentent de transformer les Paces en « portails santé » et les antennes Paces en « mineures santé » sans aucune autre modification qu'un changement de nom, la réforme aura échoué, ce qui serait très dommageable. Notons, et c'est un point positif de ce projet de loi, que le Gouvernement, en supprimant les épreuves classantes nationales, signe la fin de trois ans de bachotage intensif. Pour accéder au troisième cycle, les étudiants devront désormais avoir une note minimale à des examens qui resteront nationaux et valider les acquis du deuxième cycle par des simulations et des oraux. La commission de la culture, de l'éducation et de la communication a également souhaité que les études de santé prennent mieux en compte les questions d'implantation territoriale des futurs professionnels de santé et, en particulier, que les étudiants en médecine de deuxième et troisième cycles se voient offrir des stages en zones sous-denses. Enfin, il nous a semblé indispensable que ces mêmes étudiants bénéficient de programmes d'échanges internationaux, aujourd'hui sous-développés dans le cursus des études de santé, en particulier en médecine.

Gouvernement, vous l'aurez compris, est contraint d'aller vite. La réforme de la première année des études de santé l'oblige à publier les décrets d'application de la loi avant la rentrée prochaine pour que les étudiants puissent s'informer, notamment à travers Parcoursup.

qui, à terme, ne peut que fragiliser un projet de loi pourtant à même de créer les conditions d'une stratégie globale tant attendue. Mes collègues et moi-même resterons donc très attentifs à la mise en oeuvre de cette réforme pour faire en sorte que les objectifs poursuivis se concrétisent réellement. La parole est

les inégalités territoriales d'accès aux soins minent la cohésion nationale et notre pacte social en ajoutant une nouvelle fracture sanitaire et sociale aux nombreuses fractures, qu'elles soient territoriales, numériques, économiques ou en matière de transports, qui traversent déjà notre pays. Dans ce contexte, et en cohérence avec l'attention constante qu'elle porte à la problématique des déserts médicaux depuis sa création, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable s'est saisie pour avis du projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé, en particulier des dispositions du texte ayant des conséquences territoriales et de celles relatives à l'intégration du numérique dans notre système de soins. À cet égard, j'observe avec regret que les constats posés dans le rapport de 2013 du président Hervé Maurey ou dans mon rapport pour avis de 2015 sur le projet de loi de modernisation de notre système de santé sont toujours d'actualité.

Aussi, lors de la présentation de mon rapport pour avis, la majorité des membres de la commission, toutes sensibilités politiques confondues, a tenu à rappeler son attachement au principe d'égal accès aux soins, corollaire du droit à la santé défini par le préambule de la Constitution de 1946, et à la mise en oeuvre de mesures de bon sens pour mieux réguler la répartition des professionnels de santé sur l'ensemble de notre territoire. Malgré l'accélération du rythme d'adoption des lois relatives à la santé depuis dix ans, les inégalités d'accès aux soins se creusent sur l'ensemble du territoire et les défauts de notre système de soins demeurent les mêmes, à savoir un cloisonnement entre médecine de ville et hôpital et une difficulté à assurer un parcours de soins continu pour l'ensemble de nos concitoyens. Si toutes les professions de santé sont concernées, les inégalités d'accès aux médecins sont particulièrement marquées, alors même qu'ils occupent une place centrale dans notre système de santé avec leur rôle de prescripteur. Les écarts de densité entre départements varient de 1 à 3 pour les médecins généralistes et de 1 à 8 pour les spécialistes, voire autour de 1 à 20 pour certaines spécialités comme la pédiatrie ou la gynécologie, avec des disparités infradépartementales encore plus fortes. Ces inégalités vont continuer de se renforcer dans les années à venir, car la densité médicale retrouvera son niveau de 2015 seulement à horizon de 2030. D'ici à 2025, près d'un médecin généraliste sur quatre aura cessé d'exercer. Il ne faut pas sous-estimer les conséquences de cette situation sur la santé des populations, car la carte des déserts médicaux se superpose à celle de la mortalité précoce, comme le montrent plusieurs géographes de la santé. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas Qui plus est, les inégalités d'accès aux soins pèsent sur les finances publiques pour un montant estimé entre 900 millions et 3 milliards d'euros par an par la Cour des comptes. Par ailleurs, les dépenses de santé et de médicaments sont plus importantes là où la densité de médecins est forte, sans que l'état de santé des populations concernées justifie cet écart. Réguler l'offre de soins, c'est non seulement améliorer l'accès aux soins de nos concitoyens, mais aussi maîtriser l'évolution des dépenses de santé. Au cours de mes auditions, dont certaines ont été menées avec le rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, notre collègue Laurent Lafon, que je salue, la grande majorité des personnes et organismes que j'ai pu rencontrer ont exprimé des doutes sur la capacité du projet de loi que nous examinons à améliorer à court terme le quotidien de nos concitoyens. Ainsi, la réforme du n'aura qu'un effet limité, voire aucun effet, sur la répartition des futurs professionnels de santé sur le territoire. Du reste, je constate un recours important à des ordonnances sur des sujets aussi sensibles que les hôpitaux de proximité. En outre, plusieurs mesures me paraissent d'une portée limitée et essentiellement technique.

réguler l'offre de soins et réaffirmer le principe d'égal accès aux soins sur l'ensemble du territoire ; libérer du temps médical dans tous les territoires en allégeant les contraintes administratives pesant sur les professionnels, en développant les partages de compétences et en soutenant le déploiement de la

Aussi, avant de conclure mon propos, je souhaiterais vous poser une simple question, mesdames les ministres : quand comptez-vous prendre les décisions pragmatiques et conformes à l'intérêt général qui s'imposent pour apporter une réponse durable à l'enjeu de l'égal accès aux soins sur l'ensemble de notre territoire ? Nous passons

de santé. Face aux inégalités croissantes en matière d'accès aux soins, comment penser que l'efficience de notre système de santé passe essentiellement par une réorganisation et une mutualisation de moyens rabotés, chaque année, dans le cadre Comment ne pas dénoncer les dangers que ce projet comporte en réformant la carte hospitalière et en réduisant les hôpitaux de proximité à de véritables coquilles vides ? Alors, bien sûr, quelques mesures vont dans le bon sens, et si notre motion n'est pas votée, nous les soutiendrons. Mais elles sont noyées par votre refus de sortir du carcan de l'austérité budgétaire. Ainsi, vous proposez la suppression du que nous demandions depuis longtemps. Mais c'est une mesure en trompe-l'oeil, puisque vous en transférez la responsabilité aux présidents d'université sans leur donner plus de moyens. Et pourquoi ne pas l'avoir aussi supprimé pour les paramédicaux, singulièrement les orthophonistes, qui manquent, sur tous les territoires, en exercice libéral comme hospitalier ? En outre, ce projet de loi fait la part belle aux ordonnances, restreignant les droits du Parlement. Vous nous avez expliqué, madame la ministre, qu'il était nécessaire de faire vite pour inscrire dans Parcoursup la suppression de la Paces pour 2020. Même si nous apprécions positivement votre intention de venir nous présenter les études d'impact et les ordonnances, convenez qu'il est compliqué de vous accorder ce blanc-seing. Trente années de réformes successives, dont vous assumez la continuité, ont conduit notre système de santé dans l'impasse. Aujourd'hui, tous les voyants sont au rouge. Pour ne prendre qu'un exemple récent, mardi 28 mai, à midi, pendant cinq minutes, le président de Samu-France a appelé à cesser symboliquement le travail pour dénoncer « le point de rupture jamais atteint ». Et il a été largement suivi. Il faut décréter l'état d'urgence sanitaire dans notre pays. Trop nombreux sont nos concitoyennes et nos concitoyens à ne plus pouvoir accéder à un médecin généraliste ou à un spécialiste, dans de bonnes conditions financières, de proximité et de délai. Les personnels hospitaliers sont au bord de l'épuisement professionnel généralisé. Les élus locaux sont exclus des constructions des projets de santé. Les cas de femmes accouchant dans les ambulances se multiplient, faute de maternités de proximité. Des services sont désertés par des praticiens, qui préfèrent exercer en établissement privé où ils gagnent mieux leur vie et où ils n'ont pas les mêmes contraintes. La dette des hôpitaux a atteint les 30 milliards d'euros. Les inégalités d'accès à la médecine de ville gagnent du terrain. Les ruptures de stock de médicaments se multiplient ... Nous ne sommes pas alarmistes, mais réalistes. Si notre système de santé tient debout, c'est grâce à l'engagement sans faille des personnels. Je veux ici le souligner. Il faut donc revoir notre système de santé, ce qui nécessite de mettre en oeuvre un plan d'investissement matériel, financier et humain. Ce plan n'est pas une utopie au regard des 40 milliards d'euros trouvés par le Gouvernement quand il s'est agi de faire ce cadeau, sans contrepartie, aux grandes entreprises. C'est bien une question de choix politique ! Il faut absolument sortir du carcan financier imposé par Bruxelles et mettre en oeuvre une politique ambitieuse en matière de santé. Les propositions ne manquent pas pour y parvenir. Malheureusement, nous sommes contraints par les articles 40 et 41 de la Constitution, par le recours aux ordonnances, et par la loi de financement de la sécurité sociale. Ces propositions, qui permettraient de répondre aux besoins des populations, sont notamment en contradiction avec cette nouvelle définition en trois échelons des hôpitaux, sous couvert de gradation des soins, éloigne encore davantage les patients des infrastructures et des professionnels qualifiés, aggravant ainsi le phénomène des déserts médicaux, qui se multiplient en zones rurales et urbaines. Vous pouvez affirmer qu'il n'y aura plus de fermetures d'hôpitaux de proximité, mais vous les videz de leurs services essentiels, comme les urgences, la chirurgie ou la maternité et vous supprimez des lits. Lors de notre tour de France des hôpitaux et des Ehpad réalisé avec les collègues de mon groupe et les députés communistes, nous avons constaté, depuis quinze mois, la souffrance des personnels face à la dégradation des conditions de travail, le besoin de reconnaissance des métiers face à un sentiment d'écrasement par la machine administrative et, enfin, l'urgence d'embaucher du personnel pour arriver à soigner les malades comme il se doit. Je pense à une phrase entendue dans différents établissements visités : « Nous ne faisons plus de la qualité, mais de l'abattage. » Cette conception de l'hôpital public n'est pas la nôtre. Pour notre part, nous demandons depuis longtemps l'arrêt des fermetures de lits, de services, de maternités et d'hôpitaux, ce que le collectif Inter-Urgences, qui appelle à une journée nationale de manifestation à Paris, le 6 juin prochain, a mis en tête de ses revendications. En 2014, alors que notre groupe avait déposé une proposition de loi exigeant un moratoire sur les fermetures de services, d'établissements ou de leurs regroupements, la ministre de la santé de l'époque, Marisol Touraine, avait répondu que, contrairement à ses prédécesseurs, elle ne conduisait plus une politique de fermetures des hôpitaux.

comment comprendre que Martin Hirsch annonce la fermeture de plus d'un millier de lits en gériatrie à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris d'ici à 2024, sans que votre ministère réagisse ? Vous proposez de libérer du temps médical avec les 4 000 assistants médicaux pour les regroupements des professionnels de santé. Vous souhaitez favoriser l'exercice regroupé en maisons et centres de santé, nous disons : « Chiche les aspirations des jeunes praticiens à exercer en salariat dans des structures comme les centres de santé sont grandes. Donnons-leur les outils pour y parvenir en aidant réellement et concrètement les centres de santé à se développer. Il y a urgence à les accompagner en clarifiant le statut des professionnels exerçant dans ces centres, où les patients ont la garantie de bénéficier du tiers payant et de ne pas régler de dépassements d'honoraires, car il n'y en a pas. Nous n'opposons pas médecine hospitalière et médecine de ville. Nous reconnaissons et défendons leur indispensable complémentarité. Nous portons, avec nos collègues députés du groupe de la Gauche démocrate et républicaine, un projet alternatif de santé que nous avons élaboré avec des actrices et acteurs de notre système de santé, rencontrés tout au long de notre tour de France pour apporter une réponse immédiate aux problématiques dénoncées. Selon nous, l'urgence sanitaire nécessite d'agir tout de suite, sans attendre 2022, et de mettre en place un plan d'investissement pour une santé de qualité, accessible à toutes et à tous, financé par la suppression de la taxe sur les salaires dans les hôpitaux, par la suppression du CICE, du CIR des exonérations de cotisations patronales et par une véritable lutte contre la fraude patronale aux cotisations sociales. Avec cet argent, nous serions en capacité d'améliorer l'accès aux soins en créant 100 000 emplois à l'hôpital public et de revaloriser les carrières et les rémunérations des personnels. Est-il acceptable que les salaires des infirmières et des infirmiers en France soient les plus bas de tous les pays développés, selon l'OCDE ? Avec cet argent, il est aussi possible de revenir sur les groupements hospitaliers de territoire, de créer 100 000 emplois statutaires par an, pendant trois ans, dans les filières gériatriques et les Ehpad, de revaloriser le point des conventions collectives du secteur d'aide à domicile, d'instaurer une véritable démocratie sanitaire en remplaçant les agences régionales de santé par des conseils cantonaux de santé, et en substituant aux conseils de surveillance des hôpitaux des conseils d'administration avec un droit de veto pour les représentants des personnels et les élus locaux. Avec cet argent, il est possible de mettre en place un pôle public du médicament pour retrouver notre souveraineté en matière de production en France et de revaloriser le secteur psychiatrique pour garantir la continuité et la proximité du soin relationnel. Bref, je n'entre pas dans le détail de nos 86 propositions. Il ne s'agit pas d'une liste à la Prévert, mais d'une réorientation des recettes de la sécurité sociale vers une autre politique de la santé. C'est une question de choix politique. Nous regrettons, madame la ministre, que votre gouvernement s'inscrive dans la continuité des précédentes lois en matière de santé- loi HPST, dite loi Bachelot, et la loi Touraine. Comment comprendre cet entêtement à poursuivre et à aggraver une politique qui a échoué et qui nous conduit aujourd'hui à la situation de pénurie de médecins, de recrudescence des renoncements aux soins et à la souffrance des personnels qui peut déboucher sur des sur des drames ? Cette politique ayant prouvé son inefficacité, il faut en changer, et ce de fond en comble. Ce n'est malheureusement pas ce que vous faites avec ce projet de loi. Mes chers collègues, écoutez-nous, écoutez les infirmières de Valence qui chantent : « Y a de la colère dans les cathéters ! » Écoutez les personnels des urgences qui se mobilisent sur tous les territoires de notre pays. Votez notre motion tendant à opposer

je mets fin au suspense : nous ne soutiendrons pas cette motion tendant à opposer la question préalable. Nous avons, nous aussi, repéré les faiblesses du projet de loi- ou plus exactement les manques

Maintenir une administration de la santé hypercentralisée et, en même temps, affirmer vouloir adapter les moyens d'action aux besoins des territoires ne nous apparaît pas opérant. Nous estimons que le projet de loi manque d'ambition. Il se limite ainsi à fixer un cadre général ce qui, avec le recours aux habitations à légiférer par ordonnance, aboutit à un texte qui manque d'épaisseur. Le Parlement ne peut donc remplir pleinement son rôle de législateur.

Alors que la santé ne figurait pas parmi les thèmes choisis par le Président de la République, la question de l'accès aux soins s'est imposée dans le grand débat national. Les Français attendent des réponses pour un meilleur accès aux soins. C'est la raison pour laquelle nous considérons que nos travaux doivent se poursuivre pour nous permettre de débattre et d'enrichir encore le texte. Le groupe Les Républicains votera contre cette motion. La parole est à M. Michel Amiel,

Le scrutin est ouvert.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

après plusieurs mois de travail avec tous les acteurs de santé, des heures d'auditions, de débats en commission des affaires sociales, et plus d'une centaine d'amendements adoptés, conformément aux règles de nos institutions, nous continuons aujourd'hui d'examiner, au sein de l'hémicycle, le projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé. Ce projet de loi est la traduction d'un engagement du Président de la République, redonner du souffle à notre système de santé ». Ma Santé 2022 constitue une réponse concrète aux besoins quotidiens des Français en matière d'accès aux soins. Ainsi, il y a consensus, me semble-t-il, sur le fait que Ma Santé 2022 reste un engagement collectif : c'est le plan de transformation tant attendu de notre système de santé, pour une meilleure organisation des professionnels au bénéfice des patients. Il s'agit, d'une part, de faire face aux inégalités dans l'accès aux soins, de plus en plus de Français rencontrant des difficultés pour accéder à un médecin dans la journée et étant parfois contraints de se rendre aux urgences par défaut. d'autre part, de donner corps aux aspirations des professionnels à mieux coopérer entre eux, à disposer de davantage de temps pour soigner leurs patients et à être formés autrement. À la lecture de ce projet de loi, on peut retenir, me semble-t-il, une dizaine de mesures phares illustrant mes propos liminaires. La plus emblématique d'entre elles est la suppression du, pour permettre la formation d'un nombre de professionnels de santé répondant aux besoins de nos territoires. Répondre à l'enjeu de la démographie médicale est indispensable pour notre pays. L'objectif est d'augmenter de 20 % environ le nombre de praticiens formés. I de ce texte vise ainsi à améliorer le parcours de formation des professionnels de santé. On y trouve la réforme du deuxième cycle des études médicales et la suppression des épreuves classantes nationales, pour une orientation tenant mieux compte des compétences et aptitudes des élèves.

À l'article 7, un nouvel échelon infrarégional en matière de programmation de l'offre sanitaire et médico-sociale sera institué au niveau législatif par la création des projets territoriaux de santé.

L'ensemble des acteurs de santé que notre groupe a auditionnés ont préconisé une meilleure synergie entre l'hôpital et la médecine de ville. Nous nous réjouissons que cet article réponde à leur recommandation. À l'article 8, avec avec notamment la création des hôpitaux de proximité pour les soins du quotidien- médecine, gériatrie et réadaptation -, il s'agit de réviser en profondeur la carte hospitalière. Les premiers hôpitaux de proximité seront labellisés en 2020, l'objectif étant d'en créer 500 à 600 d'ici à 2022. Ils sont plus que jamais nécessaires, dans un contexte de vieillissement de la population et d'augmentation des maladies chroniques. Ils assureront des missions hospitalières en médecine polyvalente : soins aux personnes âgées, soins de suite et de réadaptation, consultations de spécialités et consultations non programmées.

permettra de libérer du temps médical, pour un meilleur accès aux soins. Notre système de santé pourra s'appuyer sur de nouveaux métiers, comme ceux des assistants médicaux.

Pour conclure mon analyse de ce texte, j'évoquerai le titre III, qui répond au souhait du Gouvernement de développer le numérique en santé. Ma Santé 2022 permettra de mettre en place des outils numériques pour les patients et les professionnels : ordonnance électronique, espace numérique de santé et développement de la télésanté. Ces nouvelles technologies devraient participer à une mise en cohérence et déboucher sur de nouvelles synergies entre professionnels libéraux, hospitaliers et médico-sociaux. Il s'agira de s'assurer de la protection des données de santé de tous les Français à tous les à tous les âges de la vie. Enfin, je ne peux terminer sans évoquer les outre-mer et les enjeux de santé auxquels ils doivent faire face. Ma Santé 2022, c'est d'abord,

Notre groupe présentera plusieurs amendements visant à développer l'attractivité du territoire et à désengorger le système de santé local. C'est ensuite une faculté de médecine de plein exercice aux Antilles. La faculté de médecine des Antilles existe depuis 1988. Elle doit désormais jouer pleinement son rôle dans la formation des futurs médecins de la région. Actuellement, nos étudiants partent vers l'Hexagone à partir de la quatrième année afin de poursuivre leur parcours.

un amendement visant à améliorer le dispositif de l'article 21 en outre-mer. J'espère que vous serez, mes chers collègues, sensibles à l'appel des Ultramarins sur cette question.

Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues,

Pendant ce temps, vous faites le choix du maintien de la compression des dépenses de santé, à tel point que l'on parle aujourd'hui de cure d'austérité, alors qu'il faudrait un véritable plan d'urgence. Vous faites le choix de la rigueur plutôt que celui de l'amélioration des conditions de travail, amélioration nécessaire pour assurer la sécurité et le soin des patients. Bref, vous faites le choix de l'austérité financière plutôt que celui de

Nous proposons un plan d'urgence et de rattrapage pour l'amélioration de la formation des étudiants en médecine comprenant notamment la construction rapide des CHU pour la région parisienne et des CHR en province, le déblocage des crédits et des postes pour le développement du cycle d'enseignement et la mise en place d'un plan de construction d'urgence de lits hospitaliers publics. » Presque cinquante ans plus tard, les faits nous donnent malheureusement

et les ARS. Pour augmenter le nombre d'étudiantes et d'étudiants formés, il faut augmenter les moyens des universités consacrés à l'enseignement et les capacités d'accueil en stages, je vous avais d'ailleurs interpellée sur ce sujet, madame la ministre. Il ne faudra pas que le futur décret remplace l'évaluation par d'autres critères de sélection. Concernant les mesures pour lutter contre les déserts médicaux, vous prévoyez de favoriser le cumul emploi-retraite des médecins en diminuant les cotisations complémentaires. Sans compensation financière de l'État, une telle diminution des cotisations pourrait affecter les comptes des retraites. La commission des affaires sociales a adopté un amendement visant à exonérer les praticiens exerçant en zones sous-denses, alors qu'il existe déjà des exonérations fiscales et sociales sans effet sur l'installation. Ces nouveaux dispositifs d'incitation ne changeront rien à la situation. La priorité devrait être de revitaliser les territoires, pour les rendre attractifs pour les jeunes médecins, en y laissant les services publics que votre gouvernement supprime à tour de bras. Nous le savons, de nombreux jeunes professionnels ne souhaitent plus travailler seuls 24 heures sur 24. Ils aspirent à une vie de famille et aux loisirs, ce qui est légitime.

Concernant l'organisation de la santé dans les territoires, les GHT, les groupements hospitaliers de territoire, sont devenus, depuis leur création en 2016, des outils de restructuration hospitalière et de concentration des moyens hospitaliers, soit de véritables mastodontes au détriment des petits hôpitaux. Trop souvent, les plans de retour à l'équilibre s'enchaînent, mais les GHT ne servent qu'à partager les difficultés, sans augmentation des moyens alloués.

Votre gouvernement applique sa politique libérale à notre système de santé. Pour notre part, nous défendrons une autre logique, car la santé n'a pas de prix. La parole

D'aucuns y voient la marque d'un pragmatisme qui choisit de s'attaquer à un système de soins de moins en moins adapté aux défis sanitaires de notre temps, sans mettre en scène un débat théologique. D'autres soulignent le manque d'ambition du texte, son côté patchwork, et posent une question : cette loi est-elle de nature à apporter des réponses aux grandes questions de santé publique ? Est-elle à la hauteur des défis ? Aux uns et aux autres, l'avenir répondra.

Avec ce texte, vous procédez comme jamais à une dépossession parlementaire. Nous ne mettons pas ici en cause le principe du recours aux ordonnances, légitime lorsque technicité et concertation se conjuguent. Mais nous rejetons la prétention d'un exécutif qui s'attribue une question aussi fortement politique que la carte de l'offre de soins par la conjugaison des ordonnances prévues aux articles 8 et 9. Les hôpitaux de proximité et l'ensemble des autorisations de soins sont des sujets majeurs, politiques avant d'être réglementaires. Nous souscrivons volontiers au principe de gradation et de meilleure répartition territoriale. Mais il convient ne pas marginaliser le Parlement, ce qui irait à rebours de l'évolution politique des dernières années, la santé ayant progressivement dépassé son statut de première préoccupation personnelle des Français pour devenir un sujet de débat collectif, sociétal et politique.

Mais nous savons que c'est le second cycle qui est déterminant dans la construction des représentations professionnelles et, donc, dans le devenir des étudiants. Nous approuvons également la suppression du verrou final, les ECN, qui perturbent ce second cycle.

point. En outre, nous constatons que, sous la pression de la pénurie, les fondements de notre organisation des soins et du partage des tâches sont mis en question. Soyons clairs. Oui, le partage des tâches doit aller plus loin qu'aujourd'hui. Des professionnels de santé sont sous-valorisés et sous-utilisés, alors qu'ils ont la compétence pour mieux contribuer aux parcours de soins et mieux articuler le sanitaire et le médico-social. Il nous faut trouver le bon équilibre mieux les reconnaître et mieux prendre en compte leurs savoirs et leurs savoir-faire, sans méconnaître la nécessaire délimitation entre les fonctions de diagnostic, de soin et de délivrance des produits de santé. Le confusionnisme qui se répand ne constitue une réponse satisfaisante ni pour les professionnels ni pour les usagers. À cet égard, le texte transmis par l'Assemblée nationale n'a pas atteint un équilibre satisfaisant. Le numérique dans le domaine de la santé, riche de progrès et d'innovations, est exposé aux mêmes dérives : il est un complément, une composante utile, au parcours de soins. Mais prenons garde à ce qu'il n'engendre pas un système de soins injuste, où certains verraient un médecin en face d'eux tandis que d'autres n'auraient droit qu'à un professionnel de santé derrière un écran. Je vous laisse deviner quels habitants de quels territoires auraient accès à telle ou telle solution. La même interrogation s'applique aux origines et aux classes sociales. Le numérique n'est pas un pis-aller à la désertification médicale. Il ne doit pas être à l'origine d'une médecine à deux vitesses. Nous devons donc affronter plus volontairement la question de la désertification. Ce projet de loi, vous en conviendrez, serait entaché s'il ne marquait pas un nouveau volontarisme en la matière. Les mesures incitatives produisent des effets, mais trop lentement. au conventionnement sélectif, il produirait à coup sûr des effets collatéraux qui en feraient un remède peut-être pire que le mal. Nous avons donc proposé à nos collègues de la majorité sénatoriale et de l'ensemble des groupes, qui ont accepté, de travailler ensemble à une solution. Je salue leur ouverture et leur sagesse.

La mesure aurait un effet important et déterminant en termes d'attribution de temps médical, là où les besoins sont les plus importants, à un horizon singulièrement raccourci de trois ans. Elle est de nature à résoudre, en complément des dispositifs existants, la question qui nous est posée. Madame la ministre, sur bien des sujets, votre projet de loi ouvre des pistes intéressantes. Oui, le statut des praticiens hospitaliers, les PH, doit être réformé. Oui, nous devons mieux accueillir les praticiens à diplôme hors Union européenne. Oui, l'espace numérique de santé est un défi enthousiasmant. Nous constatons seulement que ce projet a insuffisamment mûri et qu'il gagnerait à un travail plus approfondi. Ce n'est pas un hasard si la procédure parlementaire normale prévoit deux lectures dans chaque assemblée.

Le texte qui sera adopté par le Sénat sera, nous l'espérons et nous y travaillons, amélioré. Nous nous prononcerons en fonction des résultats auxquels nous parviendrons. À vous, madame la ministre, qui nous présentez une copie bien trop blanche, et qui de ce fait transformez le vote d'une loi en une question de confiance, je voudrais dire que vos propos

Tous sans exception ont dressé un diagnostic extrêmement précis et pertinent de la situation. Je pense notamment à la loi Hôpital, patients, santé et territoires du 21 juillet 2009 ou, plus récemment, à la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016. Le bilan dressé voilà dix ans est malheureusement toujours d'actualité. Il faut bien le reconnaître, aucune de ces grandes lois n'a réussi à réformer en profondeur l'organisation de la santé dans notre pays,

est depuis longtemps reconnu pour être globalement performant et efficace, par rapport à ce qui existe chez nos voisins, il se heurte à de nombreuses difficultés et doit plus que jamais s'adapter aux enjeux actuels. Vous l'avez rappelé : « Nous sommes confrontés à un système trop cloisonné - entre ville, hôpital, médico-social, ou entre public et privé, entre professionnels de santé eux-mêmes - mettant insuffisamment en valeur la fluidité des parcours, la coordination entre professionnels, la qualité et la prévention. Par ailleurs, l'accès aux soins s'est complexifié en raison notamment de la métropolisation et de l'évolution des mentalités. Les jeunes médecins ne veulent plus exercer leur métier de la même manière que leurs prédécesseurs. Ils veulent plus de liberté et plus de loisirs, et souhaitent trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le médecin généraliste, c'était autrefois un homme et sa femme, qui était son assistante ; c'était un projet de couple.

Aussi, madame la ministre, deux questions s'imposent tout naturellement aujourd'hui : comment le texte que vous nous présentez pourra-t-il corriger les insuffisances des précédentes lois et quelles voies nouvelles explore-t-il ? Nous le savons bien, une réforme d'envergure ne peut se faire sans la mobilisation de moyens humains et financiers correspondants. Nous ne pouvons que le regretter, ce projet de loi n'aborde pas cette question pourtant essentielle.

Madame la ministre, vous connaissez l'attachement du Sénat, et tout particulièrement du RDSE, au débat parlementaire ! J'ai déjà eu l'occasion de le dire dans cet hémicycle : les ordonnances constituent une forme de législation déléguée qui affaiblit le rôle du Parlement. Et, dans le climat actuel de défiance à l'égard de nos institutions, un tel affaiblissement n'est pas souhaitable. Certes, lors de votre audition, vous vous êtes engagée à venir présenter chacune des ordonnances devant notre commission et à réaliser une étude d'impact. Mais, en définitive, vous nous privez de participer à l'écriture de dispositions importantes. Pour autant, ce texte comporte de nombreuses avancées que nous tenons à saluer. Je pense évidemment à la réforme des études médicales, et notamment à la suppression, attendue par tous, du, même si nous savons que le nombre d'étudiants admis en deuxième année dépendra en partie des capacités d'accueil des universités. auront-elles les moyens de former les 20 % supplémentaires de praticiens que vous escomptez ? Vous supprimez également la Paces, qui favorise le bachotage et déshumanise les étudiants, ainsi que les épreuves classantes nationales. C'est une très bonne chose. Les mesures proposées permettront par ailleurs de privilégier la diversité des profils et de prendre en compte, outre les connaissances des étudiants, leurs expériences et leur projet professionnel. Nous approuvons également la réforme du statut de praticien hospitalier, même si celle-ci relève, là encore, d'une ordonnance. Je me félicite toutefois de la précision apportée par notre président-rapporteur quant à l'encadrement des écarts de rémunération entre les personnels titulaires et les permettra peut-être de mieux lutter contre le recours à l'intérim médical, sujet sur lequel je vous sais, madame la ministre, particulièrement impliquée. S'agissant du volet relatif à l'organisation territoriale de la santé, nous saluons l'instauration du projet territorial de santé, qui devrait permettre une véritable coopération entre les professionnels de ville, l'hôpital et le secteur médico-social, et une meilleure coordination de l'offre de soins. Nous sommes en revanche plus circonspects au sujet des hôpitaux de proximité, conçus comme le pivot de l'offre de soins sur les territoires. Il est en effet regrettable que le projet de loi, sur un sujet aussi sensible, renvoie en grande partie à une ordonnance, d'autant que, dans nos territoires, l'inquiétude est grande. Ces hôpitaux devront renoncer à leurs plateaux techniques, ce qui signifie la fin de la chirurgie et de l'obstétrique.

que votre priorité était de tout faire pour répondre à l'angoisse de la désertification médicale, dont il faut rappeler qu'elle ne concerne pas uniquement le milieu rural. Plusieurs mesures vont dans ce sens outre la « suppression » du, vous prévoyez notamment d'étendre le dispositif de médecin adjoint aux zones sous-denses et d'attribuer de nouvelles tâches aux pharmaciens, aux infirmiers et aux sages-femmes. Si ces mesures sont satisfaisantes, certains sénateurs du RDSE déplorent l'absence de mesures permettant la régulation de l'installation des médecins dans les territoires. Nous craignons en effet que la seule incitation financière à l'installation de jeunes médecins ne suffise pas à résoudre le problème de la désertification médicale. S'agissant enfin des Padhue, la clarification des règles va dans le bon sens. Néanmoins, de par leur positionnement géographique, certains territoires de la République doivent pouvoir facilement recruter des professionnels ressortissants de pays voisins. est l'objet de l'article 21 , qui étend à la Guadeloupe et à la Martinique un dispositif existant déjà en Guyane. J'ai d'ailleurs déposé un amendement dont l'objet est son extension à mon territoire, Saint-Martin. Madame la ministre,

un encombrement des urgences par des pathologies qui devraient être traitées en médecine de ville, sans parler des problèmes de rupture d'approvisionnement en médicaments, dont le Sénat s'est saisi en juillet dernier à la demande du groupe Les Indépendants et du sénateur Jean-Pierre Decool- à ce sujet, madame la ministre, vous avez annoncé un plan d'action d'ici à la fin du mois de juin. La France a la chance d'avoir un système de santé qui compte parmi les meilleurs au monde. Nous disposons d'excellents professionnels, d'une sécurité sociale parmi les plus complètes, d'un réseau hospitalier étendu et d'une recherche médicale de pointe- en la matière,

La réforme des études contribuera, en supprimant le, à préserver nos filières médicales tout en humanisant la formation de nos médecins et en augmentant progressivement les capacités de formation de nos universités, en lien- nous l'espérons -avec les hôpitaux périphériques, les cliniques et les médecins généralistes.

paraît importante. Notre groupe défendra un amendement commun à plusieurs groupes visant à favoriser la mise à disposition par la faculté ou par les hôpitaux périphériques d'étudiants en dernière année de troisième cycle,

La création de projets territoriaux de santé vise avant tout à mieux coordonner l'offre de soins dans les territoires afin d'améliorer les parcours de soins dans l'intérêt des patients et des professionnels de santé- nous y sommes favorables. Le développement d'un réseau renforcé d'hôpitaux de proximité- c'est l'objet de l'article 8 -devrait permettre de repenser l'offre de soins à l'échelle des territoires, dans une logique de subsidiarité et de complémentarité entre médecine de ville et médecine hospitalière. Nous serons attentifs au contenu de l'ordonnance qui en précisera précisera le fonctionnement et la gouvernance. La numérisation de notre système de santé constitue un autre versant important du projet de loi. La généralisation et l'enrichissement du dossier médical partagé contribueront à améliorer la cohérence et la continuité des soins délivrés. Avec le DMP, les pharmaciens, qui sont bien répartis sur le territoire, pourront, dans le cadre de protocoles établis avec le médecin traitant, s'investir davantage dans les soins prodigués Nous regrettons la suppression par la commission du droit opposable à bénéficier d'un médecin traitant dans les déserts médicaux. Aussi notre groupe défendra-t-il un amendement pour rétablir cette disposition ; il n'est pas concevable que des Français soient pénalisés financièrement et voient leur parcours de soins dégradé faute de médecin traitant.

aux personnes ayant été victimes d'un infarctus du myocarde, en l'absence de facteur de risque de récidive. Mesdames les ministres, mes chers collègues, dans nos territoires périurbains et ruraux, nos compatriotes attendent en premier lieu de cette loi des mesures efficaces pour résoudre les problèmes

dernière année de troisième cycle de devenir médecins adjoints dans ces territoires. La mise en oeuvre de cette mesure est possible ; elle doit être organisée à partir des hôpitaux de proximité.

du texte ainsi circonscrit, nombre de nos amendements ont été déclarés irrecevables au titre de l'article 40, mais surtout de l'article 45,

Un petit rappel, au préalable : les professionnels de santé se sont toujours, dans une mesure certes variable, coordonnés entre eux, avec ou sans formalisation juridique. À cet égard, la notion d'exercice « isolé », auquel les évolutions en cours sont supposées mettre fin, constitue assez largement un mythe. mythe. Quoi qu'il en soit, l'inscription de leur activité dans un exercice coordonné est un argument décisif pour l'installation des nouvelles générations de professionnels. Les communautés professionnelles territoriales de santé, ou CPTS, de taille et de modèle très variables, s'adressent aux professionnels de santé de premier comme de second recours, ainsi qu'aux acteurs du secteur du secteur médico-social. Elles nous ont paru utiles à la prise en charge des patients complexes. La place des coordonnateurs y est majeure. Tandis que les équipes de soins primaires, ou ESP, organisées autour du premier recours et centrées sur les généralistes, visent à la prise en charge d'une patientèle, les CPTS tendent à organiser et à structurer une action sanitaire territoriale plus populationnelle. Le constat est clair : la réussite de ces initiatives tient toujours à la force de volonté et à la ténacité de leurs instigateurs, dont il faut saluer l'engagement, mais aussi au soutien apporté par les équipes locales de l'ARS, qui doivent être facilitatrices et non directives. Des bémols, néanmoins : la difficulté, parfois, à mobiliser les spécialistes, et le frein que constituait l'instabilité juridique entourant le dispositif de coordination et son financement.

L'enchevêtrement de ces dispositifs d'appui, qui fonctionnent à une échelle territoriale souvent différente de celle des CPTS, entretient un sentiment de confusion bien compréhensible chez les professionnels de santé. Certains de nos interlocuteurs se sont prononcés en faveur d'une fusion des différents dispositifs d'appui ou du pilotage des plateformes par les CPTS elles-mêmes. Mais l'essentiel est bien de développer l'idée d'un guichet unique de coordination.

Les GHT ont-ils permis de développer les relations avec la médecine de ville ? De nombreux GHT ont fait de cet objectif un axe de leur projet. Toutefois, le bilan apparaît, là aussi, inégal. Le déploiement des CPTS est attendu comme un moyen de faciliter ces échanges, mais les efforts devront également venir du monde hospitalier. Un élément indispensable à cette coopération entre médecine de ville et hôpital sera en outre le développement d'outils numériques interopérables. Pour le reste, je soutiens évidemment notre rapporteur Alain Milon et salue l'équilibre trouvé dans ses propositions.

Aucun territoire n'échappe véritablement à cette problématique qui cristallise les angoisses voire les peurs, pour ne pas dire les colères. Le manque de médecins peut tout aussi bien se ressentir s'agissant des généralistes que des spécialistes. Certains territoires cumulent ces difficultés. Dès octobre 2017, soit quatre mois seulement après votre entrée en fonction, madame la ministre, vous lanciez, aux côtés du Premier ministre, un premier plan pour renforcer l'accès territorial aux soins, preuve de votre prise de conscience précoce sur cette question primordiale d'aménagement des territoires. En septembre dernier, le Président de la République présentait sa stratégie de transformation Ma santé 2022. Ce plan de réorganisation de notre système était largement salué, notamment par les professionnels de santé, qui y voyaient la traduction de votre engagement à rechercher des solutions concrètes. Le projet de loi Santé, que nous examinons aujourd'hui, ne représente qu'un chapitre de ce plan. Il vise à réformer les études des futurs professionnels de santé, en supprimant notamment le, à réorganiser notre système de santé afin de libérer du temps médical et de structurer les territoires, et à créer une véritable plateforme des données de santé. Il suscitera néanmoins beaucoup d'impatience et d'insatisfaction, car il ne répondra pas immédiatement aux difficultés d'accès aux soins. Le recours à de nombreuses ordonnances est également une source d'inquiétude. Un seul exemple : la labellisation des hôpitaux de proximité, dont la définition et la gouvernance restent encore assez floues, suscitera forcément soit le bonheur soit l'exaspération des élus et des professionnels d'un territoire.

Aussi avons-nous identifié trois pistes essentielles qui seront traduites, pour partie, en amendements visant à regagner du temps médical et à implanter les futurs médecins sur les territoires.

Cessons de concentrer nos étudiants dans les grandes métropoles- ils y restent souvent une fois leurs études terminées. Certains territoires donnent l'exemple : Laval accueillera à la rentrée prochaine des cours retransmis de la faculté d'Angers. Cette proposition ne peut se traduire par un amendement ; son sort dépendra de la volonté des universités et de leurs doyens. Merci à vous, mesdames les ministres, de les intéresser à une telle ouverture priorité aux stages. Nous le savons : les stages ambulatoires sont un levier essentiel pour faire découvrir les réalités des territoires fragiles, pour promouvoir la richesse des modes d'exercice et pour orienter les vocations des étudiants. J'identifie plusieurs conditions pour faire de ces stages des expériences réussies, donnant envie de s'installer durablement dans ces territoires : offrir aux étudiants de bonnes conditions matérielles, et ce dès les stages d'externat garantir la qualité de l'encadrement et diversifier les lieux de stage, ce qui implique de mieux prendre en compte les retours d'expérience des stagiaires et de faciliter l'agrément des maîtres de stage- nous proposerons des amendements en ce sens organiser des politiques d'accueil des étudiants dans ces territoires, non seulement par la promotion du cadre de vie, mais aussi par la rencontre avec le réseau des professionnels de santé desdits territoires. Troisième piste : favoriser le partage des tâches. Le profil type du médecin d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Les 80 heures par semaine en pratique isolée sont derrière nous

Avec le vieillissement de la population et le développement des maladies chroniques, nos concitoyens doivent se rendre régulièrement chez leur médecin traitant ou chez un spécialiste. C'est pourquoi nous devons favoriser le partage des tâches et regagner du temps médical.

Il est également nécessaire de fluidifier les parcours des professionnels de santé, en facilitant les exercices mixtes- c'est d'ailleurs ce que vous proposez, madame la ministre. Dans la continuité de vos propositions, nous voulons autoriser la pratique d'une activité libérale aux praticiens salariés à temps plein des Espic, dont l'adoption aurait pour effet de permettre un meilleur partage des tâches, tout en restant très vigilante sur la nécessité de maintenir un haut niveau de qualité des soins. L'objectif n'est pas de déléguer à tout va- cela mettrait en danger à la fois les professionnels et les patients. propos, je souhaite vous livrer un témoignage. Déléguée à l'accès aux soins avec le député Thomas Mesnier et le docteur Sophie Augros, j'ai pu mesurer, au cours de nos déplacements, combien le dialogue et l'accompagnement étaient nécessaires et essentiels. Expliquer les dispositifs, rencontrer les acteurs, relever les difficultés, comprendre les enjeux liés à chaque territoire, mettre du lien entre institutions et professionnels : autant d'actions qui mériteraient une véritable structuration. Or, sur les territoires, la déclinaison des mesures est perfectible. Nos concitoyens, les élus et les professionnels eux-mêmes ont besoin de mesurer les effets de la politique nationale. Il convient de communiquer au plus près du terrain pour fédérer tous les acteurs. Je pense toutefois qu'un effort de simplification et de clarification est nécessaire et permettra une meilleure adhésion. Je suis persuadée par ailleurs que les élus locaux ont un grand rôle à jouer- vous l'avez dit, madame la ministre -, à la condition qu'ils maîtrisent pleinement l'ensemble des dispositifs. dispositifs. Si ce projet de loi suscite globalement l'enthousiasme des Français, d'après un sondage publié aujourd'hui par un grand quotidien national, ceux-ci demandent aussi des mesures coercitives.

Dessiner le paysage de demain, en matière de santé, est indispensable ; quant à vos ambitions, madame la ministre, nous les partageons toutes, tous autant que nous sommes. Mais je crois beaucoup, au-delà d'un projet de loi, à la pédagogie et au partage des responsabilités pour engager une véritable dynamique.

C'est un texte administratif, qui continue de donner un pouvoir trop important, à mon sens, aux agences régionales de santé, sentiment d'autant plus marqué vu la taille XXL Nous sommes à un moment clé, madame la ministre. Ce texte arrive en discussion au Sénat après le grand débat national- cela a déjà été dit -, pendant lequel l'accès aux soins a été au coeur du débat politique, alors que le Président de la République n'avait pas retenu le sujet de la santé parmi les grands thèmes de cette

Après avoir beaucoup parlé des MSP, on ne parle désormais que de CPTS et de PTS ! Je m'exprime volontairement avec ces acronymes, comme si tout cela allait régler les problèmes d'accès aux soins.

situant entre 20 000 et 100 000 habitants, nous n'avons vraiment pas le même sens de la proximité- il faudra de la souplesse quant à leur périmètre. Tous les médecins qui exercent ont un réseau, même si ce réseau n'est pas formalisé. Mon sentiment est qu'aujourd'hui, tous ces médecins qui exercent en dehors des MSP ou qui ne seraient pas impliqués dans une CPTS ne sont plus dans vos radars, alors qu'ils soignent chaque jour des patients. Et, si la question des hôpitaux de proximité est majeure, si l'interaction entre l'hôpital et les professionnels de ville est un vrai sujet, commençons par améliorer les sorties d'hôpital Je crains que l'on ne soit en train de détricoter la médecine libérale, et je ne suis pas sûre que les solutions proposées dans ce texte pour répondre à la question de la démographie médicale aient été discutées en amont avec les professionnels. Car, si la réforme des études est une bonne chose, elle ne règle pas la question de l'installation des jeunes médecins, qui est bien au coeur des préoccupations de tous. À titre personnel, et comme vous, je suis défavorable aux mesures coercitives. Les mesures incitatives, souvent critiquées comme « ne marchant pas », ont au moins le mérite de permettre l'installation de jeunes praticiens.

Dans ce contexte, je vous proposerai, madame la ministre, comme plusieurs de mes collègues appartenant à différents groupes politiques de cette assemblée, un amendement visant à instaurer une formation professionnalisante cette proposition est le fruit ; afin de répondre efficacement aux besoins de médecins, nous proposerons que les étudiants de dernière année de troisième cycle de médecine effectuent une année de pratique ambulatoire en autonomie dans les zones sous-dotées.

Vous en conviendrez, madame la ministre, mes chers collègues, cette proposition constitue une réponse rapide, efficiente et pragmatique aux difficultés rencontrées. Cette solution viendrait parfaitement compléter la fin du, qui, elle, produira ses premiers effets sur le temps long. Je proposerai un autre amendement tendant à rendre obligatoires deux stages en médecine ambulatoire pour tout étudiant de troisième cycle. Madame la ministre, vous connaissez les vertus de la Haute Assemblée en matière d'écoute, de propositions et de défense de l'intérêt général. Je vous demande donc, dans les circonstances qu'à l'ordinaire, de vous appuyer sur l'expérience et la connaissance du terrain des parlementaires que nous sommes. Soyez à l'écoute du Sénat ! Je pense que le sujet est trop grave pour se prêter à des querelles stériles. Dans ses, le général de Gaulle évoquait la « certaine idée de la France » qu'il se faisait. Cette conception particulière de notre pays sera d'ailleurs réutilisée à maintes reprises par ses successeurs. Madame la ministre, je vous le dis très solennellement aujourd'hui : au Sénat, dans ce lieu de défense des territoires et de la proximité, nous nous ferons toujours une certaine idée de la santé.

Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, si l'annonce du plan Ma santé 2022 avait suscité un large consensus, sa traduction législative, à travers une question centrale- ces mesures concourent-elles à un meilleur accès à des soins de qualité ? -, interroge, interpelle et soulève, du fait du recours aux ordonnances, de fortes oppositions. Il y a une interrogation sur la superposition et la complexité des outils d'exercice coordonné. La volonté de mettre en réseau les professionnels d'un territoire pour organiser la prise en charge de tous les habitants et la cohérence entre des niveaux de coordination clinique, territoriale, complexe pour les cas difficiles, doivent se traduire dans des cadres juridiques souples, à la main des professionnels, pour leur permettre de s'en saisir facilement, de l'adapter aux besoins locaux, en ayant l'assurance de financements pérennes. doute sur le lien entre proximité et efficacité dans l'évolution souhaitée des GHT. J'insiste sur trois points de vigilance. D'abord, il faut que les nouvelles synergies permettent bien aux établissements périphériques de bénéficier des ressources médicales de l'établissement support pour garantir leur attractivité le rôle, maintenu ou non, en matière de qualité et de sécurité des soins pour les commissions médicales d'établissement ? Enfin, le rendez-vous de la loi de financement posera la question cruciale de la situation financière des hôpitaux. Dans le contexte de la grève actuelle des urgences, comment demander aux personnels de s'investir dans un projet de transformation si aucune réponse n'est apportée à leur problème de court terme ? forte opposition quand le Gouvernement, par le biais des articles 8, 9 et 10, se prépare à redessiner par ordonnance la carte de l'offre de soins hospitalière sur l'ensemble de la France. Les autorisations sont « le trésor de guerre des hôpitaux », m'expliquait récemment un chef d'établissement, d'autant plus dans un contexte de grandes inégalités territoriales. Madame la ministre, vous vous engagez à un travail de concertation. Mais c'est dans la discussion parlementaire que les élus doivent définir précisément les critères et règles d'une nouvelle organisation. Mes chers collègues, les membres du groupe socialiste et républicain sont résolument engagés dans la lutte contre les « déserts médicaux ». Après avoir formulé de nombreuses propositions, parce qu'il s'agit de l'intérêt général et parce que l'urgence est de répondre aux demandes de nos concitoyens désemparés, nous sommes totalement partie prenante d'une démarche commune,

En juin 2018, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie évoquait une « crise majeure d'un système touché dans toutes ses composantes ». Il invitait à « reconsidérer explicitement ce système de valeurs et de principes ». J'insiste sur les termes « valeurs » et « principes ». C'est leur réaffirmation qui conduira à la construction d'un système de santé conjuguant égalité, efficacité, innovation et solidarité, en mesure de répondre aux énormes besoins de santé des territoires. La parole

Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, voilà plus d'un an, le Premier ministre nous annonçait vouloir mettre fin aux « rafistolages en santé ». Cette volonté s'est ensuite traduite avec la présentation, au mois de septembre 2018, du plan Ma santé 2022. Avec ce projet de loi, vous ajoutez une pierre à l'édifice bancal qu'est ce plan. Madame la ministre, ce texte était attendu par les patients, par les professionnels de santé et par les étudiants en médecine, médecine, car le diagnostic est grave et partagé par tous, y compris sur ces travées. Si notre système de santé est aujourd'hui à bout de souffle, les Français sont, eux, tout simplement à bout. Chacun dans cet hémicycle est en effet confronté dans son territoire à l'une de ces situations : manque de moyens financiers pour un hôpital, manque de personnels soignants ou encore développement de zones en voie de désertification médicale. Il n'est pas anodin que la question de l'accès aux soins se soit imposée lors du grand débat national. De nombreux citoyens renoncent aux soins faute de professionnels disponibles. Annoncé comme une « transformation du système de santé », ce texte ne traite pas de plusieurs sujets essentiels, comme la prévention ou la revalorisation et l'attractivité des professions de santé libérales et hospitalières. rien non plus sur la recherche et l'innovation, alors même que la compétitivité de la France se dégrade dans le domaine pharmaceutique. Madame la ministre, que le Parlement ne soit pas pleinement associé à cette réforme. En effet, le projet de loi comporte de trop nombreuses mesures qui relèvent de futures ordonnances, comme les hôpitaux de proximité. Nous voilà privés d'un débat qui aurait pu enrichir le texte grâce à nos expériences dans les territoires, notre connaissance du terrain, des établissements et des besoins. Toutefois, ce projet de loi comporte tout de même quelques points positifs qu'il faut souligner, comme la réforme du statut de praticien hospitalier et la création de l'espace numérique de santé. Mais plusieurs dispositions nous interrogent. Si la suppression du et la refonte des premiers cycles des études vont dans le bon sens, qu'en est-il de l'accueil des nouveaux effectifs ? Qu'est-il prévu pour que les universités s'adaptent à l'arrivée de nouveaux élèves alors que la plupart des amphithéâtres sont déjà saturés ? Même question pour l'accueil de nouveaux internes dans les hôpitaux. Comment être certain que la suppression du profitera aux déserts médicaux, alors que moins de 15 % des étudiants en médecine choisissent le secteur libéral et qu'il n'est absolument pas souhaitable d'envisager des mesures coercitives d'installation ? Le maillage du territoire et la coordination entre acteurs sont nécessaires pour répondre au mieux aux situations de désertification médicale. Veillons à ne pas suradministrer la santé. Laissons se développer les initiatives locales. Laissons les professionnels s'organiser Ce projet de loi est donc un début de réponse aux maux dont souffre notre système de santé. S'il contient quelques avancées, il n'est pas assez ambitieux. Et nous déplorons encore une fois

pour travailler avec vous et faire avancer le texte dans le bon sens, afin qu'il améliore le quotidien des patients et des professionnels de santé. La

essentiellement sur des disciplines scientifiques et technologiques. Dès lors, il ne faut pas s'étonner que nos jeunes médecins aient envie de travailler dans les CHU les plus performants avec de la technologie de pointe, au détriment

de décloisonner, de permettre plus de liberté d'organisation pour que les territoires puissent répondre aux besoins et rendre l'exercice médical et paramédical plus attractif dans les déserts médicaux. À mon sens, la réponse, c'est ce projet de loi.

s'agit d'être en appui des territoires les plus fragiles et de répondre aux demandes des jeunes médecins qui cherchent aujourd'hui un exercice salarié. Nous souhaitons libérer du temps médical. C'est l'objet des assistants médicaux. Nous espérons évidemment que la convention médicale sera signée le 15 juin prochain. Le volet télémédecine va permettre de mieux orienter les patients. Il ne joue pas un rôle supplétif ; il s'agit vraiment de faire gagner du temps dans l'exercice médical pour orienter les malades qui en ont vraiment besoin vers des soins de recours.

dégelé l'intégralité des réserves et des crédits mis en réserve, soit 415 millions d'euros- cela faisait de très nombreuses années que l'intégralité du dégel n'avait pas été rendue aux hôpitaux publics. Une nouvelle délégation budgétaire de 300 millions d'euros est intervenue en mars 2019. Nous avons augmenté de 0,2 % les tarifs d'hospitaliers c'est la plus forte hausse des tarifs hospitaliers depuis dix ans. Nous avons mis dans la balance 200 millions d'euros pour le financement de la qualité des soins dans les établissements de santé. Nous avons annoncé 100 millions d'euros de mesures nouvelles pour la psychiatrie, renouvelés chaque année. Nous avons ajouté 50 millions d'euros pour les soins de suite

La métropolisation est un phénomène international. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a annoncé qu'il manquait d'ores et déjà 12 millions de professionnels de santé dans le monde. Par conséquent, sauf à repenser nos organisations, nous ne sommes pas en mesure, aujourd'hui, d'attirer ou de former en l'espace de quelques années un nombre de médecins suffisant pour compenser les manques. Cela nécessite

miser sur des incitations financières ou des exonérations fiscales pour les médecins. Aujourd'hui, les médecins souhaitent s'installer dans des territoires où leur exercice professionnel est attractif. C'est ce que nous faisons avec les maisons de santé, les centres de santé pluriprofessionnels, l'augmentation des postes de médecins salariés- répond à leur demande -, la possibilité de cumul emploi-retraite pour les médecins les plus âgés, les statuts mixtes entre la médecine de ville et la médecine hospitalière ... Tout cela contribue à rendre l'exercice médical plus attractif. Monsieur Jomier,

Une mobilisation des ARS pour leur faire connaître les outils est absolument nécessaire. Je compte aussi sur les associations d'élus pour mieux informer les élus locaux de tous les outils dont ils peuvent se saisir. également sur les mesures coercitives. Pour que des mesures coercitives fonctionnent, il faut qu'il y ait un nombre suffisant de professionnels à répartir sur un territoire donné. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Seules des organisations innovantes seront en mesure de répondre aux besoins.

aux acteurs le pouvoir de s'organiser et aux ARS le soin de les accompagner. Ce n'est pas du tout un texte administratif ou normatif. Vous soulignez aussi que le thème de la santé n'avait pas été choisi par le Président de la République lors du grand lors du grand débat national. C'est tout à fait normal. Nous avions déjà travaillé avec tous les acteurs dans le cadre d'une large concertation qui a duré plus de six mois. Le texte était en cours de rédaction présenté aux parlementaires dès le mois de mars à l'Assemblée nationale. Il était logique que le grand débat national nous alimente sur des mesures de santé qui auraient pu figurer en plus dans la loi. Nous avons regardé ce qui était proposé. Il s'agissait essentiellement de constats,

En d'autres termes, nous n'avons pas pensé que la santé n'était pas prioritaire ; nous avions d'ores et déjà travaillé à la rendre plus équitable sur le territoire grâce à ce projet de loi.

Cette double exigence trouve sa concrétisation dans le besoin d'une démocratie sanitaire renouvelée, plus large, avec davantage de pouvoirs et de contre-pouvoirs pour les représentants du personnel, les usagers et les élus.

concertation préalable à l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale sur le juste équilibre entre impératif d'efficience économique, qualité de soins et qualité de vie au travail. Il existe déjà une structure consultative, la Conférence nationale de santé, placée auprès du ministre chargé de la santé, dont la mission consiste justement à faire vivre la concertation et les réflexions autour des questions de santé. Ce « Parlement de la santé » de 120 membres représente les collectivités territoriales, les usagers du système de santé, les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, les organisations syndicales et patronales, les acteurs de la cohésion et de la protection sociales, les acteurs de la prévention, les offreurs de services de santé et les représentants des organismes de recherche, des industries des produits de santé et des personnalités qualifiées. Il est saisi pour avis sur les projets de loi de santé publique comme celui dont nous discutons actuellement, mais il n'est malheureusement pas sollicité concernant les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Vous me répondrez, madame la ministre, que notre groupe insiste sur les finances,

Cela n'a pas eu de conséquences sur le texte, non plus que notre opposition au Sénat. Nous sommes donc parfaitement conscients que cet amendement ne suffira pas à instaurer une véritable démocratie sanitaire, mais son adoption serait un pas positif dans cette direction. Quel est l'avis de la

d'organiser une concertation chaque année portant spécifiquement sur le thème évoqué par Mme Gréaume. On pourrait tout à fait envisager que la Conférence nationale de santé travaille de manière ponctuelle sur cette question dans le cadre d'une proposition ou d'un avis. Il ne me semble cependant pas opportun d'y affecter chaque année une large part des moyens de la Conférence nationale de santé alors que d'autres thèmes relatifs à la santé publique méritent tout autant de faire l'objet d'une concertation. En outre, l'article 10 A

Le titre I vise tout d'abord à réformer la formation des professionnels de santé. Trois moments clés sont visés : l'entrée dans les études de santé- c'est l'objet de l'article 1 -, l'entrée dans le troisième cycle de médecine et le choix d'une spécialité- c'est l'article 2 -et la formation continue des professionnels de santé- c'est l'article 3. Si les nouvelles orientations proposées recueillent le consensus des acteurs, elles ne constitueront pas le coeur des réformes qui seront mises en place. Les trois premiers articles se bornent en effet à l'affirmation de grands principes dont la traduction concrète est renvoyée à la voie réglementaire ou à l'ordonnance. Nous devons donc croire sur parole le Gouvernement quant aux modalités effectives de la réorganisation des études de santé. Comme je l'ai souligné, la communication gouvernementale autour de ces mesures apparaît pourtant partiellement trompeuse, et je crains que la réforme des études de santé ne fasse au total de nombreux déçus. Sur ce premier volet, la commission des affaires sociales a choisi de ne pas retenir les propositions visant à inscrire le contenu de certaines parties de la formation des professionnels de santé dans la loi.

Le titre I comprend par ailleurs des mesures éparses touchant à l'organisation des carrières en santé. On y trouve notamment un toilettage du CESP et un élargissement de l'exercice en tant que médecin adjoint. La principale mesure est portée par l'article 6, qui vise à réformer l'emploi hospitalier. Sur ma proposition, la commission des affaires sociales a complété ce titre par des mesures constituant constituant une incitation forte à l'ancrage rapide des jeunes médecins dans un territoire et auprès d'une patientèle. L'article 4 prévoit ainsi que ceux qui s'installeront dès la fin de leurs études bénéficieront d'une large exonération de cotisations sociales, quel que soit leur mode d'installation. Nous avons, dans le même temps et en conséquence, souhaité limiter l'exercice en remplacement à une période de trois ans sur l'ensemble de la carrière des médecins diplômés.

défavorables aux amendements visant au renforcement des dispositifs d'exercice alternatif à l'installation : la multiplication de ces outils pourrait au total avoir des effets délétères sur l'installation pérenne de médecins dans un territoire de santé. La

sera sans doute l'un des plus emblématiques de ce projet de loi, l'un des plus médiatisés également. Et pour cause, il correspond à une urgence : former plus de médecins pour faire face à la baisse démographique et répondre aux besoins de santé sur tous les territoires, même si ses effets ne se font sentir que dans dix ans. Vous vous étonnez, madame la ministre, que tous les pays du G7 vivent la même pénurie de médecins, mais tous les pays du G7 mènent la même politique libérale et l'amplifient ! C'est une mauvaise politique qu'il faut changer. à opposer la question préalable, qui a été rejetée. Vous acceptez enfin de supprimer le, ce qui va dans le bon sens. Avec les syndicats, nous dénonçons depuis longtemps ce couperet, convaincus que ce mode de sélection, d'une part, est responsable de la pénurie de professionnels de santé que nous connaissons actuellement et, d'autre part, que la première année commune aux études de santé, la Paces, constitue un véritable cauchemar pour les étudiants, et un gâchis d'intelligence et de compétences. Cette ultra-sélection, synonyme d'échec pour 75 % des étudiants,

en fonction d'objectifs nationaux pluriannuels établis par l'État et sans moyens supplémentaires. Comment pensez-vous, mesdames les ministres, que les universités pourront accueillir et former plus d'étudiants en médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie dans ces conditions ? En fait, il s'agit d'une proposition somme toute limitée, puisqu'elle permettra, selon vous, madame la ministre, une augmentation maximale de 20 % des effectifs, même si j'ai bien compris que vous ne teniez pas à ce que l'on rappelle ces chiffres. Je crains qu'il ne s'agisse donc plutôt d'un desserrement du, comme cela se pratique depuis quelques années, et d'une régionalisation de ce. Une fois de plus, vous restez au milieu du gué. Enfin, je ne saurais terminer mon propos sans souligner que la diversification des profils et des parcours est une mesure positive, à même de favoriser une prise en charge plus humaine des patients, ce que nous soutiendrons sans réserve ! La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly,

pour former les futurs médecins afin de justifier l'instauration de la sélection dans les études de médecine. L'argument des moyens matériels et des places de stage avait été invoqué pour limiter le nombre d'étudiants. À l'époque déjà, les parlementaires communistes dénonçaient une pratique qui consiste à créer la pénurie pour mieux justifier les mesures d'élimination. Ils demandaient une augmentation constante et prolongée du nombre des étudiants à former. Malheureusement, pour former, il aurait fallu se donner davantage de moyens financiers

faudra déployer, que vous le vouliez ou non, madame la ministre, des moyens supplémentaires ! Or nous sommes très inquiets quand nous entendons le Président de la République annoncer que le système restera sélectif et dire qu'il n'est pas question de rogner sur l'excellence de la formation. En

Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, alors que la pénurie de médecins contraint plus de 5 millions de nos concitoyens à vivre dans un désert médical, nous ne formons pas assez de futurs professionnels. Le système est tel qu'un grand nombre de jeunes sont éjectés de la formation médicale cours des deux premières années d'études. Si la disparition du nous satisfait, de nombreuses interrogations demeurent. Ce sont les facultés de médecine et les ARS qui auront désormais la main sur la formation des futurs médecins, et détermineront les effectifs d'étudiants en fonction des besoins des territoires. Mais comment s'organisera la nouvelle formation ? Le seul critère de débouchés locaux ne risque-t-il pas de remettre en cause le caractère national du diplôme ? Tiendra-t-il compte de la mobilité des étudiants, en France ou à l'étranger, en fonction de leurs souhaits ou de leurs projets professionnels ? Se pose surtout la question des moyens financiers dont il faut doter les universités pour former plus et mieux. Travailleront-elles à moyens constants ou des moyens supplémentaires seront-ils engagés ? Qu'en est-il, enfin, de la question de la réforme globale des études de médecine ? La suppression du est une bonne nouvelle, mais les enjeux de la démocratisation des études médicales et de la régulation de l'installation des médecins ne sont que partiellement traités. La parole est à M. Bernard Jomier, Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, l'article 1 vise à instaurer un certain nombre de mesures auxquelles nous ne pouvons qu'être favorables. La réforme des modalités d'admission en deuxième année d'études médicales en fait partie. En effet, la suppression de la Paces de la Paces met fin à un système organisé sur l'échec des étudiants, et c'est une bonne chose. Néanmoins, j'attire l'attention du Gouvernement : il est nécessaire que les nouvelles modalités de sélection soient garantes de l'égalité des chances entre les candidats, ce que permettait l'anonymat des épreuves qui prévalait jusqu'alors. Cette notion ne doit pas disparaître de nos textes. Venons-en à la suppression du. Cette suppression serait la mesure phare permettant de répondre à la problématique de la désertification médicale. Or, si nous n'y sommes pas opposés, rien ne prouve que le nombre

Enfin, on ne peut pas donner la priorité aux capacités de formation des universités sur les besoins de santé de la population dans la détermination du nombre de professionnels à former.

des pratiques douces et plus respectueuses de leur santé. Les scandales sanitaires provoqués par certains médicaments ne sont pas étrangers à cette prise de conscience collective. La médecine par les plantes s'inscrit par ailleurs dans le désir de développement durable que nous voulons tous.

On commence tout juste à en mesurer les effets sur notre santé. N'a-t-on pas trouvé des traces d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires dans les moules et les poissons ? N'assiste-t-on pas à la féminisation des poissons ? Nous devons nous montrer à la hauteur des enjeux et

Il s'agit d'humaniser la formation de nos médecins en supprimant la forme de sélection par l'échec qui caractérise actuellement l'admission en deuxième année. Nous le savons, en Paces, l'échec s'élève des étudiants ont eu le bac S avec mention. Le système de réorientation actuel après un échec est quasi inopérant, ce qui témoigne d'un dysfonctionnement majeur, et coûteux pour les finances publiques, de cette filière particulièrement sélective. Bien sûr,

leurs formations- cela a été dit par notre rapporteur, que je suis complètement dans ce domaine -et, d'autre part, « en même temps », selon la formule consacrée, à augmenter significativement le nombre d'étudiants.

! Sachez que la rédaction de l'article 1recueille le consensus de la grande majorité des acteurs de santé, comme des acteurs de la formation.

et ce n'est pas coutume, fait une avancée remarquable en réformant le et en supprimant les épreuves classantes. Toutefois, il me semble qu'il faut aller plus loin en inscrivant dans la loi la notion de « souhaits de l'étudiant », qui tient à deux éléments. Tout d'abord, je l'ai déjà évoqué, nous assistons non pas à une réforme pure et simple du mais, finalement, à un report de son initiative. Les notions de et de capacité d'accueil comportent de nombreux points communs.

interrégionale. De fait, la prise en compte des souhaits et aspirations des étudiants dans le processus d'orientation doit permettre aux ARS et aux universités d'anticiper au mieux les volontés de mobilité et de gérer les flux d'étudiants. Cette problématique se ressent déjà dans certains centres universitaires, principalement au niveau des licences 3 et des masters, ce qui explique d'ailleurs pourquoi de nombreuses universités ont mis en place des outils de concertation en amont. Cela doit également permettre de transformer radicalement la vision de l'orientation et d'en faire non un processus par défaut, mais un processus positif. À ce titre, la mention actuelle de « projet d'études » est largement insuffisante, car ce dernier renvoie exclusivement,, à la question de l'intégration sur le marché de l'emploi. Or les choix des jeunes, lorsqu'ils avancent dans leur orientation, sont bien évidemment guidés par cette finalité, mais pas seulement. La présence, dans le corps enseignant, de tels ou tels spécialistes, la possibilité de se diriger vers tel ou tel stage, les spécialisations et options disponibles, sans compter les éléments extérieurs aux études mêmes, font que l'orientation doit s'appuyer sur les souhaits des étudiants et non se contenter de plier les aspirations des jeunes aux moyens mis en oeuvre. Quel

permettre à un jeune issu d'une zone sous-dotée de faire au moins sa « mineure santé » à proximité de chez lui pour éviter une coupure trop importante par rapport à son lieu de vie. Nous

Lafon. Comme la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable souhaite que l'exigence d'une répartition équilibrée des futurs professionnels de santé figure parmi les objectifs des études de santé.

J'attire l'attention de l'ensemble de nos collègues sur le fait que la refonte du n'aura, à elle seule, qu'un effet limité, voire aucun effet, sur la répartition des professionnels de santé sur le territoire. Qui plus est, il y a un risque de voir les moyens alloués aux universités se concentrer sur les établissements les plus importants et les plus éloignés des zones sous-denses. Pour toutes ces raisons, il me semble raisonnable de faire apparaître, dès le stade des études, la nécessité de penser la démographie médicale

comme une préoccupation majeure des citoyens dans le cadre du grand débat national destiné à répondre à la crise de défiance à laquelle votre gouvernement est confronté, madame la ministre. Nous pensons donc qu'il faut aller plus loin et faire entendre la voix des territoires. C'est en ce sens que nous avons travaillé en commission, proposant des amendements qui apportent des réponses concrètes aux habitants des zones où la présence médicale est trop faible, voire inexistante. L'article 1 du projet de loi réorganise le premier cycle des études de santé. Il nous paraît essentiel que cette réorganisation de la formation permette de mieux faire correspondre les ressources disponibles aux besoins de santé des Français rendus inquiets par la disparition des médecins généralistes et spécialistes sur leur territoire. Il est ainsi proposé de compléter l'article 1 en précisant que les études de médecine, par leur organisation, favorisent la répartition équilibrée des futurs professionnels au regard des besoins de santé. Il pourrait en effet être utile que les futurs médecins soient formés là où les besoins d'implantation sont les plus patents en adaptant étroitement la répartition des étudiants en médecine aux besoins de santé constatés. L'objet de notre amendement- qui vient en soutien de ceux qui sont défendus par les deux rapporteurs pour avis -est donc de prendre en compte, dès le stade de la formation et de l'organisation des études, une répartition équilibrée des futurs professionnels. Il s'agit d'anticiper les besoins des territoires et de lutter contre la désertification médicale le plus en amont possible.

de ces précisions. Selon moi, le premier et, à vrai dire, le seul objectif des études de santé est de former des professionnels prêts à exercer leur métier dans les meilleures conditions possible. Toujours selon moi, le but des études de médecine n'est pas non plus de répondre aux carences de l'offre de soins. Il est de former des médecins. Je me demande par ailleurs quelle serait la traduction concrète d'un tel principe. Cela signifierait-il, par exemple, que les étudiants seront assignés à la faculté de leur département d'origine ou à celle dans laquelle ils ont fait leur première inscription ? Qu'adviendrait-il s'ils souhaitaient, ensuite, suivre une spécialité qui n'est pas enseignée dans cette faculté ? Je crains en outre que, en adoptant un tel principe, nous ne posions les bases d'une formation au rabais des professionnels de santé. Si demain, nous envoyons un grand nombre d'étudiants en médecine faire des stages dans des zones en déficit de professionnels, ils ne seront pas aussi bien encadrés que ceux dont les stages se déroulent dans des zones mieux pourvues en

madame la ministre, ? Il nous semble que ce deuxième alinéa est structurant et pose de grands principes qui définissent les objectifs et le déroulement des formations.

ce qui n'est pas négligeable non plus en la matière. Bien sûr que nous formons des professionnels de santé pour ce qu'ils sont et pour répondre aux besoins de santé du pays

Les besoins sont différents d'un territoire à l'autre, on le sait déjà depuis longtemps, mais les fractures se sont aggravées sur le plan de l'accès aux soins et le nombre des professionnels formés doit clairement répondre à ces fractures et à ces besoins. Il faut

C'est tout simplement terrifiant. Compte tenu du fait qu'il n'y a eu que cent cinquante jours depuis le début de l'année, nous sommes au-delà du chiffre communément admis depuis des décennies d'une femme assassinée tous les trois jours. Comment en sommes-nous arrivés là ? Alors que les discours volontaristes se multiplient à l'envi, pourquoi n'arrivons-nous pas à résoudre ce scandale d'un autre âge ? Il faut donc agir, autant qu'on le peut et au plus près possible des femmes. Or, souvent, les médecins sont en contact avec ces femmes ; prises dans un engrenage pervers, elles ne portent pas plainte, mais elles viennent consulter pour leurs blessures. Il s'agit donc de faire en sorte que tout médecin soit sensibilisé à la fois sur les mécanismes de harcèlement moral, mais aussi sur les chiffres, les statistiques, les études sociologiques et les faits dans leur dure réalité. Cette sensibilisation doit permettre aux médecins d'agir avec tact et respect et d'accompagner ces femmes qui sont psychologiquement dans l'incapacité de regarder la réalité en face, réalité qui les met en grave danger de mort. Cela concerne bien les médecins qui doivent jouer leur rôle premier, soigner les blessures physiques et psychiques, mais aussi

les enseignements relatifs aux violences faites aux femmes, aux stéréotypes de genre et au respect du corps d'autrui font partie intégrante des programmes de formation des médecins, notamment dans le module « Vulnérabilité »

c'est un idéal qui nous anime. La médecine scolaire est un levier puissant pour cela, puisqu'elle permet un accès automatique aux soins et un suivi des enfants. Or la médecine scolaire n'est plus en mesure de remplir sa mission. En quelques années, nous sommes passés de 57 % à 47 % d'enfants qui ont passé la visite obligatoire à 6 ans. Cette diminution est d'autant plus préoccupante que le projet de loi pour une école de la confiance abaisse l'âge de l'instruction obligatoire de 6 ans à 3 ans.

Quel est l'avis de la commission ? Il me paraîtrait peu équitable d'inscrire dans la loi un objectif de promotion spécifique de la médecine scolaire. En outre, la mise en place d'actions de renforcement de l'attractivité de la médecine scolaire et des autres spécialités en difficulté me paraît plutôt relever de l'accompagnement des étudiants organisé par chaque université. La commission a donc émis un avis défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement

dans certaines facultés. Ainsi, certains établissements pourraient proposer moins de places qu'auparavant. Je sais que ce n'est pas votre objectif, madame la ministre, mais c'est pourtant une conséquence envisageable pour les universités qui ont, ces dernières années, augmenté leur nombre de places en Paces. Et même s'il faut avoir une vision nationale de la suppression du, nous pensons que les calculs du ministère de l'enseignement supérieur sont inférieurs aux besoins et que le budget actuel pour le redoublement de la Paces ne suffira pas. Ainsi, les universités et les ARS s'appuieront, pour déterminer leur, sur les capacités de formation des établissements et, on peut l'anticiper, les possibilités de stage. Notre amendement revient en fait à passer d'une logique de moyens à une logique de finalité.

la procédure relative à la détermination des objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle des formations en médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique. Le projet de loi prévoit que les universités déterminent annuellement les capacités d'accueil

qui tiennent compte des capacités de formation et des besoins de santé du territoire. Ces derniers sont eux-mêmes définis au regard d'objectifs nationaux pluriannuels établis par l'État pour répondre aux besoins du système de santé et pour réduire les inégalités d'accès aux soins. soins. Pour respecter l'autonomie des universités et instaurer une confiance mutuelle entre universités et agences régionales de santé, un avis simple des ARS est tout à fait pertinent pour répondre aux objectifs du projet de loi et il permet de prévenir d'éventuelles situations de blocage. L'amendement : La parole est à M. Vincent Segouin. Cet amendement vise à associer les acteurs de terrain que sont les URPS, les fédérations hospitalières et les conseils départementaux dans la détermination des capacités d'accueil des formations sur le territoire. La détermination des capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années sera dévolue aux universités sur la base des objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle de ces formations arrêtés sur avis conforme des agences régionales régionales de santé. Parce qu'il est important que la logique de décloisonnement entre la ville et l'hôpital intègre la réflexion dès les études médicales et parce qu'il est urgent que les universités et les ARS prennent en compte les besoins de terrains de stage en médecine de ville, cet amendement vise à faire participer les URPS et les fédérations hospitalières à la définition de ces objectifs pluriannuels. Il est également impératif que les élus départementaux soient consultés en tant que représentants politiques de la population locale, car ils ont, depuis de nombreuses années, financé ils ont, depuis de nombreuses années, financé des projets favorisant l'installation de médecins sur les territoires. L'échelon départemental, associé aux URPS, est un relais d'information absolument nécessaire à la bonne évaluation des objectifs pluriannuels. Quel

de la capacité d'accueil de l'université dans la définition des objectifs pluriannuels d'admission en deuxième cycle. Les objectifs pluriannuels d'admission en deuxième cycle constituent l'outil qui remplacera demain le. Ils doivent Ils doivent donc prendre en compte les capacités de formation des universités, mais aussi des éléments prospectifs quant aux besoins de santé de demain dans l'intérêt des patients comme des futurs professionnels. De ce point de vue, la formulation proposée n'a pas choqué la commission des affaires sociales, qui a donné un avis de sagesse.

il me paraîtrait curieux de ne pas prendre en compte les capacités de formation, et donc les moyens universitaires, pour la détermination du nouvelle version. J'espère d'ailleurs que cette prise en compte permettra, le cas échéant, d'adapter à la hausse les moyens des facultés- plusieurs responsables universitaires nous ont fait part de leur forte inquiétude face à la réforme à venir. La commission a émis un avis défavorable.

Cela ne me paraît pas une bonne idée de laisser une telle autonomie aux universités, dans la mesure où ce seront les ARS, et non les universités, qui consulteront les acteurs de santé du territoire au travers des CRSA.

par la quatrième phrase de l'alinéa 3, qui prévoit la consultation des CRSA qui rassemblent l'ensemble des acteurs cités. Il paraîtrait étrange d'ajouter à cette consultation générale la consultation spécifique de ces instances, dont je ne doute pas que l'avis sera cependant pris en compte- Mme la ministre pourra cependant nous confirmer

l'avis du Gouvernement ? Concernant l'amendement n° 734 rectifié, l'article 1 prévoit bien que l'université doit prendre en compte les objectifs

c'est pourquoi nous avons prévu un avis conforme, et pas un avis simple. Un avis conforme ne remet aucunement en cause le principe d'autonomie des universités.

la consultation des conférences régionales de la santé et de l'autonomie est prévue dans la loi ; y sont associés les URPS, les conseils départementaux, les représentants des usagers et les fédérations hospitalières.

Jean-Marie Morisset. Pour mieux définir les objectifs de formation, il est nécessaire de mieux en appréhender les besoins. L'organisation de la formation doit se faire au plus près des lieux d'exercice, sur la base d'un diagnostic partagé par l'ensemble des acteurs. Les objectifs de formation devraient être évalués en fonction de l'ensemble des lieux de stage universitaires et non universitaires et des demandes des territoires en effectifs et en compétences. Cet amendement donc à intégrer ces besoins au moyen d'une méthodologie adaptée permettant de faire remonter les besoins des établissements qui sont représentés au sein des comités régionaux de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé, ces derniers étant plus à même d'évaluer les besoins en formation.

des objectifs régionaux de formation doit prendre en compte « l'évolution prévisionnelle des effectifs et des compétences des acteurs de santé du territoire ». Il ne paraît donc pas utile de le préciser de nouveau à l'échelon national, d'autant que l'échelon territorial est plus adapté à un suivi de cette évolution.

pour leur substituer la consultation d'un organisme compétent uniquement en matière de démographie des professions de santé. La détermination des effectifs des soignants de demain ne doit pas uniquement dépendre de projections techniques liées aux professionnels les collectivités locales, les établissements hospitaliers, les représentants des patients, pour ne citer qu'eux, doivent également pouvoir donner leur avis. Sans doute le fonctionnement des CRSA n'est-il pas toujours optimal, mais ce n'est pas en les contournant

à celle des cadres. Tout cela fait de la France l'un des mauvais élèves des pays de l'Union européenne. Se pose dès lors la question des raisons d'un tel phénomène. Les conditions matérielles de vie, mais également les conditions de travail peuvent conduire à des prévalences supérieures en matière de maladies chroniques et de troubles physiques divers, notamment musculo-squelettiques. Il faut aussi reconnaître le rôle des pratiques sociales dans certains des troubles de santé que connaissent les ménages les plus précaires.

Je vois mal comment un tel objectif pourrait être pris en compte pour la détermination du nombre de professionnels à former. on peut concevoir que les inégalités territoriales d'accès aux soins soient directement liées aux effectifs de professionnels de santé- surtout à leur répartition sur le territoire

Jean-Marie Morisset. Il s'agit de mentionner explicitement dans la loi les territoires sur lesquels doit porter l'effort prioritaire de réduction des inégalités d'accès aux soins, que sont les territoires périurbains, ruraux, de montagne, insulaires et ultramarins.

La précision que tend à apporter cet amendement a été supprimée par la commission des affaires sociales, qui a considéré qu'il revenait au Sénat de veiller à la préservation de la qualité et de la concision de la loi. Outre que la précision n'apporte rien sur le plan juridique, toute énumération de ce type présente le risque d'oublier certains éléments pourtant potentiellement concernés., par exemple, des territoires urbains

des étudiants. C'est pourquoi il est proposé de permettre aux établissements de santé privés de conventionner avec les universités pour mettre à disposition leur expertise et leur savoir-faire médical et chirurgical dans le cadre des formations des étudiants. l'amendement n° 172 rectifié. L'accès aux soins, notamment l'accès à une offre médicale équilibrée et de qualité sur l'ensemble des territoires, constitue l'un des principaux enjeux de la transformation de notre système de santé. La suppression du national au profit d'une régulation territoriale devrait permettre de répondre d'une manière mieux ajustée aux futurs besoins en santé de la population. Toutefois, tous les acteurs de santé doivent être mobilisés autour de cet enjeu, tant sur la réduction des inégalités d'accès aux soins que sur l'insertion professionnelle des étudiants. C'est pourquoi il est nécessaire que les établissements de santé privés participent eux aussi à cet objectif commun. Une meilleure connaissance par les futurs médecins de l'ensemble des environnements de soins, publics comme privés, améliorera l'efficience du système et favorisera les coopérations et les équilibres sur les territoires.

L'accès aux soins, notamment l'accès à une offre médicale équilibrée et de qualité sur l'ensemble des territoires, constitue l'un des principaux enjeux de la transformation de notre système de santé. La suppression du national au profit d'une régulation territoriale devrait permettre de répondre d'une manière mieux ajustée aux futurs besoins en santé de la population. tous les acteurs de santé doivent être mobilisés autour de cet enjeu, tant sur la réduction des inégalités d'accès aux soins que sur l'insertion professionnelle des étudiants. C'est pourquoi il est proposé de permettre aux établissements de santé privés de conventionner avec les universités pour mettre à disposition leur expertise et leur savoir-faire médical et chirurgical dans le cadre des formations des étudiants. Le conventionnement porte aussi sur les conditions d'accueil. Une meilleure connaissance par les futurs médecins de l'ensemble des environnements de soins, publics comme privés, améliorera l'efficience du système et favorisera les coopérations et les équilibres sur les territoires. Quel

La rédaction ne prévoit d'ailleurs ni la portée de cette précision ni son éventuelle sanction en cas de non-prise en compte de ces besoins de formation. Deuxièmement, un tel dispositif serait en porte-à-faux par rapport à la logique proposée par l'alinéa 3 pour la définition des effectifs d'étudiants en filières MMOP.

lesquelles comprennent des représentants des établissements de santé. Il me paraît donc à la fois superfétatoire et illogique de contourner cette architecture pour prévoir une forme de consultation parallèle des seuls établissements de santé. Troisièmement, le texte adopté par la commission prévoit que la fixation des objectifs pluriannuels doit tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs et des compétences des acteurs de santé des territoires, ce qui me paraît satisfaire assez largement la préoccupation exprimée. un argument de forme et de préservation de la qualité de la loi qui vient s'ajouter à ces raisons de fond -, la rédaction proposée n'a pas sa place à cet endroit du texte, puisque l'article 1 prévoit les grands principes structurants du premier cycle des filières de santé.

pluriannuels participe aux diverses dispositions nationales prises depuis de nombreuses années pour tenter de pallier la pénurie de médecins. Il est désormais indispensable, face aux difficultés rencontrées par la population, mais aussi par les élus locaux sur tous les territoires, d'avoir une vision globale de l'ensemble des dispositifs nationaux de lutte contre la désertification médicale, notamment dans le cadre d'un « jaune budgétaire » spécifique. Quel

les seuls parcours possibles seront les licences et les classes préparatoires. Il n'est pas souhaitable de remplacer tout ou partie de l'actuel premier cycle par un cycle de licence dite « santé », qui risquerait de se traduire par une dilution de l'apprentissage des compétences, par l'impossibilité d'un enseignement professionnel au contact des patients et, par conséquent, par un allongement de la durée des études pour garantir que les compétences des futurs diplômés soient au moins équivalentes à celles que confère la formation actuelle. Les études de médecine sont indissociables de la pratique clinique. Quel est l'avis de la commission médecine. Quel est l'avis de la commission ? entendus- pour ne pas dire l'intégralité -sont tombés d'accord pour ne pas inscrire le portail santé dans la loi, car ils craignent- à juste titre, me semble-t-il -la recréation d'une nouvelle Paces sous un nouveau nom, en tout cas la mise en place d'une voie royale pour l'accès aux études de santé, en contradiction avec l'objectif de diversification des parcours prévus à l'article 1.

-pourront se faire dans des universités, y compris dans celles qui n'ont pas de facultés de médecine. Il est très important que celles-ci puissent organiser leur premier cycle de façon à permettre aux étudiants de démarrer ces formations

parce que les facultés de médecine et les doyens des facultés de médecine ont une très longue habitude de travailler ensemble pour définir qui les formations de préparation aux

entre les facultés de médecine et les universités, qu'elles contiennent ou pas des facultés de médecine, permet de répondre à cet objectif. C'est à l'issue de ce processus et sur la base des propositions qui seront formulées que seront

alors qu'une réforme permettra à des étudiants n'ayant pas eu d'enseignement dans le domaine de la santé d'accéder en deuxième année de MMOP, il est demandé aux infirmiers diplômés d'État deux ans d'exercice supplémentaires et la validation pour reprendre leurs études au même stade. Cet amendement a donc pour objet de prévoir que les étudiants en soins infirmiers aient désormais la possibilité de s'orienter vers des études de médecine dès leur deuxième année d'études, au même titre que les autres professions de santé. Puisque le projet de loi créée des passerelles nombreuses vers les études de médecine, il paraît incohérent que les étudiants en soins infirmiers continuent à devoir justifier de deux années de pratique professionnelle après l'obtention de leur diplôme pour rejoindre une formation de premier cycle en médecine.

de l'article 1, qui organise les quatre filières MMOP et la circulation entre ces quatre filières uniquement. On peut imaginer que cela peut s'arranger dans le temps ... Ensuite, la préoccupation que vous exprimez légitimement a été en partie satisfaite à l'Assemblée nationale par l'adoption d'un dispositif expérimental organisant une transversalité entre les différentes formations médicales et paramédicales : c'est l'objet des alinéas 19 à 22 de l'article 1. Sans doute cette expérimentation permettra-t-elle d'envisager le développement de passerelles entre ces différentes formations. Enfin, il ne me paraîtrait pas équitable

ce qui risquerait de déséquilibrer les chances des différents candidats en défaveur de ceux qui n'auraient pas été inscrits dans les formations d'infirmiers. La formulation

la concertation est encore en cours avec les facultés de médecine ; il y aura probablement une première liste d'admissibilité, pour éviter de faire passer plus de 50 000 étudiants à l'oral Nous devons nous prononcer sur une procédure claire. Or l'article L. 631-1 du code de l'éducation, tel qu'il est actuellement rédigé, précise qu'un « arrêté détermine les critères de répartition de ce nombre de façon à garantir l'égalité des chances

Il ne me paraît pas opportun d'y ajouter un objectif général d'égalité des chances des candidats alors qu'aucune des dispositions figurant à l'article 1 ne le traduit concrètement. Qui plus est, l'égalité des chances constitue un enjeu